du groupe d'amitié Royaume-Uni-France, issus de la Chambre des Communes et de la Chambre des Lords, conduite par Stephen Crabb. Ils sont accompagnés par notre collègue Jean-François Rapin, vice-président du groupe interparlementaire d'amitié France-Royaume-Uni. Arrivée en fin de matinée, la délégation s'est entretenue avec note collègue Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes, qui copréside le groupe de suivi sur le retrait du Royaume-Uni et la refondation de l'Union européenne. la délégation participera à un débat sur les conséquences du Brexit pour les entreprises, organisé conjointement par le groupe d'amitié et la délégation aux entreprises. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de réaffirmer les liens historiques forts qui unissent nos deux pays. La France et le Royaume-Uni doivent oeuvrer pour conserver d'excellentes relations et agir dans leur intérêt commun. Le Sénat est particulièrement attaché au dialogue interparlementaire avec le Parlement britannique, auquel il souhaite témoigner sa fidèle amitié. Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter, en votre nom à tous, à nos homologues du Parlement britannique, la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour.

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé

souhaite vous dire ma profonde satisfaction de voir les deux assemblées parlementaires aboutir à une rédaction commune sur un texte important, appelé à structurer notre système de santé pour plusieurs années. Au terme de nos travaux, le projet de loi, qui comportait initialement 23 articles, en compte 63 ; 28 d'entre eux avaient été adoptés par le Sénat dans une rédaction conforme à celle de l'Assemblée nationale ou moyennant de simples ajustements rédactionnels. Au cours de la commission mixte paritaire, 31 articles ont été adoptés dans la rédaction issue du Sénat, avec parfois quelques aménagements formels ; 14 articles insérés par notre assemblée ont été maintenus. Certes, le texte adopté par la CMP n'est pas parfait les défauts du projet de loi initial, déjà largement soulignés, n'ont pas disparu. Le texte opère toujours un renvoi que nous jugeons bien trop large au décret et aux ordonnances il constitue sur plusieurs sujets majeurs, comme la réforme du statut des personnels hospitaliers ou les évolutions de la carte hospitalière, un simple cadre d'orientations, voire une forme de « chèque en blanc » au Gouvernement. De surcroît, il laisse de côté les enjeux majeurs de la gouvernance et, selon moi surtout, du financement de notre système de santé. Je n'y reviens pas, car nous avons déjà largement évoqué ces éléments lors de nos discussions de première lecture. Nous resterons vigilants quant aux moyens qui seront déployés pour accompagner la mise en oeuvre de ce texte : c'est bien ce qui signera ou non la réussite de la nouvelle loi Santé, la troisième en dix ans. Ces réserves étant dites, je me félicite de ce que l'esprit constructif dans lequel notre assemblée avait souhaité travailler ait été partagé par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Thomas Mesnier, et, plus généralement, par l'ensemble des membres de la À l'heure où la demande d'accès aux soins se fait de plus en plus urgente dans nos territoires et où nous pouvons tous constater la souffrance des personnels hospitaliers, il aurait été dramatique de ne pas nous accorder sur la volonté de répondre à ces difficultés. Je suis très satisfait, en particulier, que le texte adopté par la commission mixte paritaire prenne largement en compte les préoccupations exprimées par le Sénat sur deux sujets majeurs l'amélioration de l'offre de soins dans les territoires et l'accompagnement de la transformation numérique de notre système de santé. Sur le premier volet, nous sommes parvenus à un accord sur une disposition emblématique de l'article 2 introduite en séance publique par le Sénat : la mise en place d'une professionnalisation de la dernière année d'internat de médecine, sous la forme d'une année de pratique ambulatoire en autonomie se déroulant en priorité dans les zones sous-dotées. Cette disposition résultait d'une démarche transpartisane portée par nos collègues Corinne Imbert, Yves Daudigny et Daniel Chasseing. Elle visait à répondre à l'attente immense que nous entendons tous dans nos territoires et qui s'est largement exprimée lors du grand débat national.

Je dois dire que l'accord auquel nous sommes parvenus en CMP a fait l'objet d'âpres négociations avec la majorité de l'Assemblée nationale comme avec les représentants des internes en médecine, concernés au premier chef. À mon sens, la rédaction retenue permet à la fois de proposer une première réponse efficace et pragmatique à l'urgence territoriale, dans un horizon temporel accessible et acceptable, et de prendre en compte les inquiétudes légitimement exprimées par les étudiants quant à la qualité de leur formation. Le dispositif adopté prévoit de systématiser le stage ambulatoire en soins premiers en autonomie supervisée, ou Saspas, pour les étudiants de dernière année de médecine générale, en l'ouvrant aux étudiants d'autres spécialités. spécialités. Si le Saspas existe depuis 2004, cette expérience de pratique ambulatoire n'est pas suivie par l'ensemble des étudiants en médecine générale, notamment en raison du manque de maîtres de stage. Ce stage, désormais obligatoire et généralisé, devra avoir une durée d'au moins un semestre- semestre- douze mois auraient été encore mieux. Tout à fait ! Dans l'organisation actuelle du troisième cycle, cela permettra aux étudiants de se succéder sur un même terrain de stage semestre après semestre, ces terrains de stage devant être prioritairement définis dans les zones sous-dotées. sera effectué sous le régime de l'autonomie supervisée. Ses contours seront définis par un décret, qui pourra notamment ouvrir la possibilité d'une supervision à distance, afin de laisser davantage de souplesse dans l'organisation des terrains de stage.

Ce stage obligatoire permettra à l'ensemble d'une promotion, c'est-à-dire près de 3 500 étudiants, de découvrir l'exercice ambulatoire dans les territoires, puis d'y poursuivre- pourquoi pas ? -son exercice professionnel. Surtout, il permettra de déployer dans deux ans l'ensemble d'une promotion sur les territoires. Ainsi, ces derniers disposeront du renfort d'étudiants parvenus presque au terme de leur formation. Cette disposition laisse en suspens la question de l'alignement de la formation de médecine générale sur celle des autres spécialités. Il me semble que la réflexion sur la mise en place d'une quatrième année en médecine générale devra être poursuivie. Le volet territorial du texte contient également une invitation des partenaires conventionnels à ouvrir des négociations sur les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins. Cette disposition, introduite au Sénat sur l'initiative de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, me semble un signal positif, d'autant qu'elle ne restreint pas la palette des outils qui pourront être déployés pour atteindre ce but. Sur le volet numérique, les enrichissements substantiels du projet de loi opérés par le Sénat ont été conservés. L'ouverture de l'espace numérique de santé et du dossier médical partagé, leviers de la coordination indispensable des parcours de soins, sera donc automatique. donc automatique. Pour éviter un retard qui pourrait ensuite être impossible à rattraper, notre assemblée avait également souhaité renforcer les exigences d'interopérabilité applicables au secteur en instituant un mécanisme de certification accompagné d'instruments à visée incitative pour les éditeurs : je pour les éditeurs : je me félicite de le voir figurer dans le texte que nous nous apprêtons à voter. Bien entendu, j'ai également quelques regrets. Nous n'avons pu maintenir certaines propositions sénatoriales qui nous paraissaient importantes. Je pense notamment à la composition des commissions médicales des groupements hospitaliers de territoires, les fameux GHT : le Sénat avait souhaité qu'elles émanent des commissions médicales des établissements parties, pour qu'elles ne deviennent pas des instances hors-sol, ou au sein desquelles les établissements supports seraient parfois les seuls représentés. Madame la ministre, nous comptons sur vous pour veiller à ce que l'application de la loi et les ordonnances qui suivront sur ce sujet préservent un équilibre entre les établissements supports et les établissements périphériques dans le cadre de l'acte II des GHT. Je regrette également que nous n'ayons pu tomber d'accord sur l'intégration dans la procédure de qualification de l'article 21 des praticiens les Ehpad. L'ambition de régler l'ensemble des cas d'ici à 2021 ne pourra être satisfaite si nous commençons par exclure une partie des praticiens contribuant au bon fonctionnement de notre système de santé, d'autant que, pour ce qui concerne les Padhue, la plupart des acteurs ont agi aux frontières de l'illégalité. Contrairement aux annonces gouvernementales, nous devrions donc entendre de nouveau parler des Padhue au cours des prochaines années. Enfin, nous avons accepté de supprimer certaines des dispositions introduites par le Sénat au regard des engagements pris par le Gouvernement. Il en est ainsi des mesures incitatives à l'installation rapide des jeunes médecins dans nos territoires : nous suivrons avec attention les mesures que vous nous proposerez dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Plus généralement, nous nous veillerons à ce que le contenu des nombreuses ordonnances prévues par le texte corresponde bien aux orientations présentées dans le cadre de nos débats. Pour ce qui concerne l'organisation de la santé au sein des territoires, nous avons insisté sur la nécessaire souplesse dans les démarches de structuration des acteurs, pour prendre en compte la diversité des situations locales. Un projet revenant à faire entrer tous les territoires dans un même moule est voué à l'échec. l'échec. Blaise Pascal l'a exprimé mieux que moi par ces mots : « La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion ; l'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. sous le bénéfice de ces observations, je vous invite à adopter le texte issu des travaux de la CMP ainsi que l'amendement de coordination qui sera présenté par le Gouvernement. Très bien

c'est une grande satisfaction lorsque les deux chambres du Parlement aboutissent à un texte commun. Une satisfaction renforcée s'agissant de ce projet de loi, car, chacun le sait sur ces travées, il y a urgence à réformer notre système de santé. Cette loi permettra ainsi, avec les autres volets de « Ma santé 2022 », de nous armer face aux nombreux défis auxquels nous devons faire face, et de garantir une offre de soins égale et de qualité pour tous. Elle nous permettra aussi de répondre aux inquiétudes légitimes des Français, aux sollicitations des élus et aux aspirations des professionnels de santé, tout aussi légitimes. Les attentes sur les territoires sont très fortes et nous devons rapidement mettre en oeuvre la loi pour que les résultats soient visibles. Si le changement de paradigme engagé autour du projet Ma santé 2022 porte déjà ses fruits, puisque les professionnels de santé libéraux ont signé les accords avec avec l'assurance maladie sur le déploiement des assistants médicaux et le financement des communautés professionnelles territoriales de santé, il nous faut maintenant traduire concrètement ces avancées pour nos concitoyens. La première orientation de Ma santé 2022 est de construire le système autour du patient, et c'est bien l'usager qui sera l'évaluateur de notre réussite. Mesdames, messieurs les sénateurs, les débats au Parlement ont été riches. Ils ont permis d'améliorer plusieurs dispositions, de lever certaines craintes et de répondre au mieux aux situations des territoires. J'aimerais revenir quelques instants sur les apports sénatoriaux retenus lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Je pense d'abord à l'article visant à fusionner les multiples dispositifs d'aide à la coordination des parcours des patients qui coexistent aujourd'hui

Je pense également à la question du numérique en santé. Vous avez initié une avancée très importante en prévoyant l'ouverture automatique du dossier médical partagé pour tous dès 2021 et l'interopérabilité des systèmes, qui fait aujourd'hui défaut sur le terrain. terrain. Je souhaiterais aussi saluer l'équilibre qui a été trouvé à l'article 2 concernant le développement des stages d'internes en médecine de ville. plusieurs d'entre vous étaient très attachés à cette disposition et je suis heureuse qu'un compromis ait pu être trouvé pour maintenir une formation encadrée tout au long des études. Loin des mesures coercitives, le texte obligera aussi les universités et les services de l'État à trouver des terrains de stage en priorité dans les territoires en tension. Ce projet de loi prépare les futurs soignants aux besoins du système de santé de demain : nous aurons désormais des professionnels de santé mieux sélectionnés, aux profils variés et davantage formés à travailler ensemble. Dans le même temps, nous créons sur tous les territoires un collectif de soins au service des patients et nous offrons aux professionnels de santé les outils pour se rassembler et coopérer. L'accord trouvé par la commission mixte paritaire porte un message fort de l'ensemble des forces politiques. Les deux chambres parlementaires ont été déterminées à répondre indépendamment des clivages partisans aux inquiétudes de nos concitoyens concernant l'accès aux soins dans tous les territoires. Mesdames, messieurs les sénateurs, je conclurai mon intervention par une note plus personnelle, car j'aimerais vous remercier des échanges sincères et éclairés que nous avons eus en audition, dans cet hémicycle ou en dehors. La question de la santé et de l'accès aux soins charrie beaucoup d'expériences personnelles, et je pense que chacun a pu exprimer ses convictions sur ce sujet. Nous nous devons à présent de réussir. Je vous remercie d'avoir donné votre accord pour engager la transformation du système de santé que nous proposons. La parole

ne va absolument pas régler les problèmes que connaît notre système de soins, singulièrement l'hôpital public. Alors que les personnels et les praticiens dénoncent leurs conditions de travail, les patients leurs difficultés quant à l'accès aux soins, les élus et les usagers l'absence de prise en compte de leurs avis dans les décisions des établissements, vous poursuivez dans la même logique que vos prédécesseurs : limiter les dépenses publiques. C'est une réponse qui a prouvé son inefficacité ou plutôt sa nocivité, plongeant notre système de santé dans une crise profonde. Madame la ministre, vous n'entendez pas la colère des professionnels, vous refusez de prendre en compte les propositions de notre groupe, qui, pourtant, sont de nature à redonner à notre système de santé les moyens de fonctionner. Aujourd'hui, ce sont 205 services des urgences sur 524 qui sont en grève dans notre pays pour réclamer des effectifs en personnels pluridisciplinaires supplémentaires, des lits d'aval nécessaires pour atteindre l'objectif « zéro patient sur les brancards » et une revalorisation des salaires de 300 euros. Travailler dans de bonnes conditions pour une meilleure prise en charge des patients, quoi de plus normal ? Or, madame la ministre, vous avez décidé avec Bercy qu'il n'y aurait pas d'augmentation des effectifs. Vous avez donc cherché des solutions ailleurs, en dégageant du temps médical pour les praticiens avec les délégations de tâches et la création des auxiliaires médicaux. Ces mesures pourraient être efficaces si la situation de l'hôpital n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. Vous sous-estimez totalement les réalités de terrain. Après des années de suppression de postes à l'hôpital, les équipes sont épuisées et n'arrivent plus à répondre aux missions qui sont les leurs. Alors que les personnels se mobilisent contre la détérioration des conditions de prise en charge des patients et de leurs conditions de travail, votre gouvernement fait adopter un amendement au projet de loi de transformation de la fonction publique pour étendre le recours aux contrats temporaires et saisonniers dans les hôpitaux. Le secrétaire d'État Olivier Dussopt ne connaît visiblement rien à la fonction publique hospitalière : il tient des propos mensongers qui me conduisent à faire un rappel au règlement. des personnels qui n'en peuvent plus, vous faites le choix de la précarisation à outrance : ils jugeront ! Vous proposez également de réorganiser les hôpitaux en trois niveaux, pour éviter soi-disant que les patientes et les patients restent plusieurs heures sur un brancard. Vous vous vantez de labelliser deux fois plus d'hôpitaux de proximité, mais cela signifie en réalité deux fois plus d'hôpitaux qui ne réaliseront plus d'activités de chirurgie ou d'obstétrique, pour ne citer que ces deux exemples. Sous prétexte que les hôpitaux de proximité manquent de praticiens, vous préférez acter la carence et les amputer de leurs principales missions. Ce faisant, d'une part, vous accélérez le phénomène de concentration de l'expertise et des moyens financiers dans les grandes structures hospitalières des métropoles au détriment des zones rurales et périurbaines ; d'autre part, vous éloignez les services de soins des habitants. À l'inverse de ce que vous prévoyez de faire avec votre loi, il est indispensable de maintenir, sur notre territoire, un maillage d'hôpitaux de proximité disposant chacun d'un service des urgences, d'un service de médecine, de chirurgie, d'une unité obstétrique, de soins de suite et de structures pour les personnes âgées, le tout en liaison avec la médecine de ville et le réseau de centres de santé, ainsi qu'avec la psychiatrie de secteur. Pour y parvenir, il faut notamment embaucher, donc rendre plus attractive la fonction publique hospitalière. La gradation des soins n'a de sens selon nous que si le premier niveau est le plus complet possible et accessible au plus grand nombre. L'accord trouvé entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et la majorité du Sénat sur la désertification médicale illustre l'importance de ne pas transformer les hôpitaux de proximité en coquilles vides. En obligeant les étudiantes et les étudiants à effectuer six mois de stage pour leur troisième et dernière année d'internat dans un territoire sous-doté, vous faites un premier pas dans la bonne direction. Mais ces 3 500 étudiants devront trouver des médecins maîtres de stages pour exercer dans les déserts médicaux. Or les maîtres de stages vont préférer choisir les hôpitaux spécialisés où se situent les services d'urgences, de maternité et de gériatrie plutôt que les hôpitaux de proximité tels que vous les concevez. En outre, nous savons toutes et tous que les étudiants souhaitent majoritairement exercer la médecine dans des structures collectives, type centre de santé, pour avoir une activité salariée. Nous déplorons que la commission mixte paritaire ait supprimé notre amendement qui visait à mettre fin à l'exercice non salarié dans les centres de santé. Votre avis de sagesse aurait mérité plus d'engagement de votre part, madame la ministre, afin que, peut-être, les députés de votre majorité nous suivent. Par ailleurs, comment ne pas évoquer le scénario antidémocratique et contraire aux droits des femmes qui s'est joué pour faire retoquer l'amendement qui avait été adopté pour allonger le délai légal de l'IVG ? Enfin, notre déception est profonde concernant les praticiens à diplôme hors Union européenne, notamment pour celles et ceux qui disposent de la nationalité française. Le Sénat avait adopté l'élargissement de l'exercice des Padhue dans le secteur médico-social, sur lequel est revenue la commission mixte du médico-social à la précarité du travail illégal et à la non-reconnaissance de leurs qualifications. Ce sont autant d'arguments qui nous conduisent à ne pas voter cette loi, d'autant qu'elle ne tire aucun enseignement de la mise en oeuvre, à marche forcée, des groupements hospitaliers de territoire et qu'elle continue d'ignorer la démocratie sanitaire. Dans son, Descartes nous invitait à douter de tout. Le moins que l'on puisse dire est que ce n'est pas la marque de fabrique de ce gouvernement. C'est fort regrettable, madame la ministre, car cela vous conduirait enfin à écouter et à entendre les professionnels de santé qui, tout comme notre groupe, ici, dans l'hémicycle, vous enjoignent à changer de politique

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons les conclusions de la commission mixte paritaire qui, le 20 juin dernier, est parvenue à un accord sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Deux voix s'exprimeront pour le groupe socialiste et républicain et, avant Nadine Grelet-Certenais, j'aborderai deux sujets. Conjuguée aux inégalités de santé- espérance de vie, prévalence de certaines pathologies dépendantes des conditions sociales ou environnementales -, la faible accessibilité aux soins d'environ 5 millions de Français, en territoires ruraux ou urbains, est l'un des facteurs les plus destructeurs de notre pacte républicain. Trois amendements initiaux portés par Corinne Imbert, Daniel Chasseing et moi-même, un travail commun où l'intérêt général et la volonté d'agir ont écrasé les rivalités partisanes, une majorité forte de 311 voix, une difficile négociation entre les deux rapporteurs- je salue l'engagement d'Alain Milon sur ce dossier -ont abouti à un vote unanime de la commission mixte paritaire sur un amendement de compromis porteur de l'essentiel, à savoir la réalisation par les étudiants de médecine générale en dernière année de troisième cycle d'un stage d'un semestre au minimum en régime d'autonomie supervisée, en priorité dans les zones sous-denses, avec une extension possible à certaines autres spécialités. Ainsi, chaque année, les étudiants en fin d'études, dans un cadre de formation réaffirmée-je pense aux remarques formulées par ces derniers -découvriront l'exercice ambulatoire dans tous les territoires, y compris dans les territoires en difficultés. Le gain en temps médical disponible pour les habitants sera immédiat. Qui soutiendra que des vocations ne naîtront pas au contact d'une réalité inégale selon les bassins d'emploi, difficile parfois sans doute, mais aussi une réalité d'abord humaine et attachante ? Bien sûr, personne ne pense que tout est réglé, mais un sillon supplémentaire a été creusé dans la lutte contre les déserts médicaux. Il témoigne de la valeur du travail parlementaire, de l'intérêt du bicamérisme, de la capacité d'initiatives du Sénat. du Sénat. Parce qu'il s'est fondé sur le seul intérêt général, il honore notre Haute Assemblée. Madame la ministre, mes chers collègues, le second point de mon propos sera d'une autre nature. Lors de la discussion, nous avions exprimé de fortes oppositions sur les articles 8, 9 et 10. Le renvoi massif à des ordonnances utilisé dans la plupart des textes examinés depuis deux ans contourne le débat démocratique et réduit à l'extrême l'apport possible des parlementaires. La notion de proximité inséparable de celle de qualité est fondamentale pour les services publics. La notion de gradation des soins est partagée. Cependant, malgré les précisions apportées à l'article 8 sur la nature des missions socles, trop d'incertitudes génératrices de craintes pour les acteurs locaux demeurent sur ce que pourrait être la future carte des hôpitaux de proximité. L'article 9 avait été voté conforme au Sénat. Le régime d'autorisations des activités de soins et des équipements lourds sera donc modifié par ordonnances. Les autorisations sont des actes essentiels dans le dessin de la carte sanitaire, « le trésor des hôpitaux » me disait un directeur d'établissement. La commission mixte paritaire a rétabli la presque totalité de l'article 10 dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, réactivant ainsi les craintes déjà formulées sur l'avenir des commissions médicales d'établissement, leur lien avec les commissions de groupement, sur la future gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. le Gouvernement se donne les moyens de dessiner à sa seule main une nouvelle carte sanitaire de notre pays, sans possibilité pour le Parlement d'en approfondir les orientations et les conséquences pour les territoires, les citoyens et les professionnels. rapidement la problématique financière. Si elle n'est pas prise en compte, la réforme ne pourra porter ses fruits. Vous devez garder, madame la ministre, une extrême vigilance sur la situation des hôpitaux, dont le mouvement des services d'urgences exprime, encore aujourd'hui, la grave instabilité. Ce n'est pas sans danger pour les patients et pour les professionnels.

du groupe socialiste et républicain sur l'article 2 de compromis ouvrant une nouvelle piste de lutte contre les déserts médicaux nous amèneront à nous abstenir sur l'ensemble du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c'est avec plaisir que je m'exprime au nom du groupe du RDSE pour la dernière étape du processus législatif de ce texte, dont nous saluons l'esprit et l'équilibre. Nous en saluons l'esprit d'abord, car il propose des outils aux mains des professionnels. Cette souplesse attendue est de bon augure pour répondre aux enjeux de la santé du XXI siècle et à la nécessaire transformation de notre système de santé. Nous en saluons également l'équilibre grâce à un compromis entre sénateurs et députés, mais aussi grâce à un débat, parfois animé, mais toujours constructif, entre des courants différents qui, d'ailleurs, s'affranchissent des lignes partisanes. Je parle, bien sûr, des désaccords qui persistent entre les tenants et les opposants de la coercition. Au sein même de notre groupe, des divergences se sont exprimées. À titre personnel, je me réjouis de l'absence de mesures coercitives dans ce texte final, grâce à l'engagement continu de la ministre et de notre rapporteur. Cette prise de position ne nous fait toutefois pas oublier l'urgence qui existe sur nos territoires et dont le Sénat s'est légitimement fait l'écho. Si les débats ont été vifs, c'est que l'inquiétude est grandissante sur cette question si centrale de l'accès aux soins. L'avenir de notre système de santé passera par des mesures fortes, qui inscrivent dans le marbre l'attachement de la France à une médecine de qualité partout et pour tous. Je crois en cette loi, car elle redit la confiance de l'État envers les professionnels de santé, dont les nouvelles aspirations sont enfin prises en compte. La coopération, d'abord, prend toute sa place dans la nouvelle organisation de notre système de santé. Nous le voyons dans nos départements, les territoires qui se portent le mieux sont ceux dont les professionnels et les élus se saisissent des outils de coordination, créant ainsi une dynamique attractive pour les jeunes qui aspirent à exercer en équipe.

J'en viens à l'article 2, qui a concentré l'essentiel des débats de la commission mixte paritaire. J'ai déjà exprimé mon désaccord sur l'introduction d'une année de professionnalisation en internat de médecine, considérant qu'elle porterait atteinte à la formation. Un accord satisfaisant a été trouvé en CMP. Sans révolutionner ni mettre en péril les exigences de l'enseignement universitaire, il inscrit dans la loi un stage de six mois, en autonomie supervisée et en médecine ambulatoire, pour les étudiants de fin de troisième cycle, ce qui les incite à se tourner davantage vers les zones en tension. Il s'agit d'un signal fort envoyé aux élus et à nos concitoyens. À charge, maintenant, pour le pouvoir réglementaire de définir l'« autonomie supervisée ». J'aimerais toutefois insister sur le fait que la question posée ici est non pas tant celle de la durée du stage ou du degré d'autonomie du stagiaire que celle de l'existence même de stages variés et formateurs en et formateurs en nombre suffisant. D'une part, les conditions requises pour l'obtention du statut de maître de stage sont si contraignantes qu'elles découragent bon nombre de médecins. Sur ce point, l'article 2 offre une première réponse, grâce à l'engagement de notre collègue Élisabeth Doineau, en assouplissant les conditions de délivrance des agréments. D'autre part, l'environnement des stages en zones sous-dotées doit également être interrogé, notamment en termes de logement et de mobilité, sans quoi ils restent inaccessibles aux étudiants. En outre, il n'est pas inutile de rappeler que les hôpitaux sont fortement dépendants des internes dans leur fonctionnement. Même si l'on considère que les formations sont encore trop « CHU-centrées », ces stages demeurent indispensables. Les études ne peuvent à elles seules être une variable d'ajustement pour compenser la carence des médecins sur les territoires. S'agissant du numérique, nous ne pouvons que saluer les avancées de cette loi, notamment les apports du Sénat conservés dans le texte final. Je citerais ainsi la généralisation de l'espace numérique de santé et du dossier médical partagé, qui permettront de centraliser les informations et les données, tout en garantissant un haut niveau de confidentialité et de sécurité. S'ils doivent bien sûr être accompagnés de garde-fous compte tenu de la sensibilité des données concernées, les apports du numérique en santé sont un enjeu majeur de notre siècle, et nous nous réjouissons qu'ils soient envisagés ainsi par le Gouvernement. Sur le même sujet, nous notons le maintien dans le texte final de notre proposition visant à adosser un plateau de télésanté à chaque hôpital de proximité. Je remercie ainsi la ministre, que nous avons réussi à convaincre du bien-fondé de cette mesure, notamment pour les patients à qui nous offrons un cadre professionnel et sécurisé pour la pratique de la télémédecine. Puisqu'il est question des hôpitaux de proximité, j'en profite pour revenir à un sujet qui a fait débat : la composition des commissions médicales d'établissement des GHT. L'Assemblée nationale a préféré renforcer la gouvernance des GHT GHT la création de commissions médicales de groupement et la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales. Sur ce point, il convient d'être pragmatique : les GHT ont vocation à assurer une continuité et une cohérence des soins hospitaliers à l'échelle d'un bassin de vie. Toutefois, l'existence d'une stratégie de groupe et d'une mutualisation plus aboutie des ressources humaines doit se faire au profit des plus petites structures, qui peinent, seules, à recruter et à fidéliser les praticiens. Il faudra veiller à ce que cette nouvelle organisation améliore la présence médicale sur tout le périmètre des GHT. Un bémol tout de même, je tiens à évoquer le cas des praticiens à diplôme hors Union européenne. Le Gouvernement ne souhaitant pas évoluer sur ce point, nous avons dû revenir en commission mixte paritaire sur les ouvertures accordées par le Sénat. Compte tenu des pénuries de médecins que connaissent certains territoires, des situations difficiles que vivent certains Padhue, mais surtout des nombreux garde-fous qui existent pour le contrôle de leurs compétences, cette loi aurait pu prévoir de plus grandes avancées, tout en conciliant qualité et sécurité des soins.

j'y tiens particulièrement, il faudra renforcer l'accompagnement de nombreux territoires que je qualifierais d'atones et pour qui la prise en main des outils législatifs est loin d'être une évidence. Pour ne pas creuser l'écart entre ces territoires et les métropoles, plus dynamiques, élus et professionnels comptent sur le soutien d'agences régionales de santé souples, aidantes et à l'écoute, afin que cette loi irrigue l'ensemble du territoire. La parole

L'un des principaux points de blocage portait sur l'article 2, plus précisément sur l'obligation, introduite par le Sénat, pour les futurs médecins généralistes de faire leur dernière année de troisième cycle « en autonomie » dans une zone sous-dotée. La commission mixte paritaire a convenu de ramener la durée à un semestre en « autonomie supervisée ». Les députés et les sénateurs ont, sur ce point, fait preuve d'un sens des responsabilités qui honore le Parlement. Alors oui, certains regretteront que leurs amendements n'intègrent pas le texte final. J'en connais quelques-uns parmi vous. Mais des compromis ont dû être concédés. J'ai moi-même renoncé à certains de mes amendements pour que, en définitive, le texte soit soutenu par le plus grand nombre, ce qui facilitera son appropriation sur les territoires. Notre responsabilité pour demain est la suivante s'emparent de l'ensemble des outils mis à disposition par ce projet de loi et de ceux qui existent déjà pour apporter des réponses concrètes à nos concitoyens. Il est question non pas de reproduire la même organisation des soins de la Bretagne à la région Occitanie, mais de donner à l'ensemble des acteurs des territoires les moyens organisationnels et techniques Les Français nous attendent sur le terrain pour construire avec les usagers, les professionnels de santé et les élus locaux un projet structuré et adapté. Nous voulons faire du sur-mesure en somme, pour gommer progressivement les inégalités territoriales dans l'accès aux soins. C'est pourquoi je me félicite de ce que perdure dans le texte final l'instauration d'une concertation au moins une fois par an entre le directeur général de l'ARS et les élus locaux sur l'organisation territoriale des soins. Dans le même esprit, les élus pourront demander à inscrire toute question à l'ordre du jour. Ils pourront, enfin, solliciter l'organisation d'une réunion spécifique lorsque les circonstances le justifieront.

Désormais, le nombre d'étudiants autorisés à passer en deuxième année sera décidé au niveau de chaque université, en liaison avec les agences régionales de santé suivant les besoins des territoires. Ensuite, nous avons convenu que la diversification et la multiplication des lieux de stage sont une priorité, si ce n'est « la » priorité. Les stages sont un levier majeur pour faire découvrir aux futurs professionnels les réalités des territoires fragiles ainsi que la richesse des modes d'exercice, et mieux orienter ainsi les vocations. Mais il n'est pas possible de développer les stages sans, dans le même temps, développer l'émergence des maîtres de stage. L'année dernière, leur nombre a augmenté de 14 %, soit 10 736 praticiens référencés. C'est important, mais il nous faut aller En termes d'organisation, l'accent est mis sur le développement des projets territoriaux de santé et des communautés professionnelles territoriales de santé. Je souscris à ces orientations, qui doivent prendre désormais leur pleine mesure. Mises à la disposition des professionnels de santé et constituées à leur initiative, ces organisations ont tous les atouts pour s'adapter au contexte local, pour structurer les liens ville-hôpital et pour fédérer les coopérations. En contrepartie d'un financement maximal de 380 000 euros, l'objectif est de faciliter l'accès à un médecin traitant et d'améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville. Rappelons que 8,6 % des Français n'ont pas de médecins traitants, les exclut du parcours de soins prévu par la loi et les prive d'un suivi régulier et adapté, ainsi que d'un meilleur remboursement des frais engagés. En complément du projet territorial, j'avais proposé que les médecins puissent être désignés conjointement médecins traitants dès lors qu'ils participent à une même communauté professionnelle territoriale de santé. La commission mixte paritaire a jugé cette mesure prématurée. J'entends l'argument. Cette proposition devra néanmoins être réévaluée lorsque les CPTS seront plus matures et auront maillé l'ensemble du territoire. Ces dernières décennies, nos dirigeants ont fortement manqué d'anticipation sur les besoins en santé des Français.

là où les professionnels sont si peu nombreux qu'ils sont trop accaparés par la patientèle, dégager un temps suffisant à consacrer à la réflexion d'une nécessaire organisation territoriale relève de l'exploit. Il faut en tenir compte et répondre à cette réalité. Si les assistants médicaux doivent d'abord permettre de libérer du temps médical, il est probable que ce temps disponible soit en définitive utilisé uniquement pour participer au travail de coordination. Dans cet esprit de réorganisation territoriale de l'offre de soins, le projet de loi crée les hôpitaux de proximité. Ils assureront le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers : médecine, gériatrie, réadaptation, entre autres. Ils n'auront cependant pas d'activité d'obstétrique ou de chirurgie, sauf dérogation. Mais la presse se fait régulièrement l'écho d'accouchements inopinés hors établissement à la suite de la fermeture d'une maternité. Madame la ministre, vous devez apporter une réponse forte à cette angoisse des jeunes et futurs parents avec le « pack maternité », qui devrait être intégré au projet Pourriez-vous envisager d'y travailler en amont avec quelques parlementaires et, éventuellement, avec le groupe-contact national que vous avez mis en place ? Les élus ont en effet de fortes attentes à cet égard. Enfin, je tiens à attirer votre attention sur deux points qui ont été rappelés par mes collègues. D'une part, malgré votre volonté d'apurer la situation des praticiens à diplôme hors Union européenne, celle-ci ne sera pas réglée pour un certain nombre d'entre eux, ce qui créera une injustice ou du moins un sentiment d'injustice qui ne peut être oublié. D'autre part, je note la désaffection significative des étudiants pour les métiers d'aide-soignant, d'infirmier, et d'autres professions du soin et de l'accompagnement des personnes âgées et handicapées. Est-ce une question de représentation ou de rémunération ? Les écoles ont actuellement beaucoup de mal à atteindre leurs objectifs, comme j'ai pu le constater en Côte-d'Or la semaine dernière. Quelques ajustements du dispositif Parcoursup seraient sans doute nécessaires. Pour conclure, je suis convaincue de la nécessité du dialogue et de l'accompagnement. Il convient de communiquer au plus près du terrain pour fédérer tous les acteurs et favoriser le partage des responsabilités afin d'imprimer une véritable dynamique. Le chantier de la réorganisation de notre système de santé passera davantage par le terrain que par la loi. Votons donc définitivement ce projet de loi et mobilisons-nous sur le terrain sur le terrain ! Madame la ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans la tribune d'honneur d'une délégation de députés du Parlement irakien, conduite par Mme Ala Talabani, présidente du groupe d'amitié Irak-France. La délégation est accueillie par le groupe d'amitié France-Irak, présidée par notre collègue Bernard Cazeau, pour une visite consacrée au rôle de la France dans la reconstruction de l'Irak. La délégation participera à un déjeuner de travail avec le groupe d'amitié, ainsi qu'à un petit-déjeuner économique avec l'Agence française de développement, la direction générale du Trésor et plusieurs entreprises françaises qui souhaitent développer leur présence en Irak. Elle sera également auditionnée par le groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens, les minorités au Moyen-Orient et les Kurdes, présidé par notre collègue Bruno Retailleau. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une intensification des relations interparlementaires, avec la perspective de la prochaine visite à l'automne du président du Parlement irakien, Mohammed al-Halboussi. La France s'est tenue aux côtés de l'Irak au sein de la coalition internationale contre Daech. Elle entend également le soutenir dans le processus de reconstruction politique et économique pour lequel le Parlement, clé de voûte des institutions irakiennes, est appelé à jouer un rôle central. Le Sénat sera attentif à toutes les sollicitations formulées par nos partenaires irakiens contribuant au renforcement des parlementarismes, garantie d'une participation inclusive de l'ensemble des citoyens à la vie politique. Mes chers collègues, permettez-moi, en votre nom à tous, de souhaiter à nos homologues du Parlement irakien la bienvenue au Sénat français ainsi qu'un fructueux séjour.

et à la transformation du système de santé. L'accord qui en résulte témoigne de la qualité du travail des deux assemblées et de la bonne volonté de chacun d'enrichir le texte sans le dégrader. Il témoigne également de l'urgence d'agir pour garantir l'accès aux soins à tous dans tous les territoires. L'amendement transpartisan, à l'article 2, que le Sénat a adopté pour professionnaliser la dernière année des études de médecine, avec un stage ambulatoire de six mois, a constitué le coeur des débats. Notre groupe se félicite du maintien de cette disposition. Plus de 45 % des médecins sont âgés de plus de 55 ans. Les départs à la retraite des généralistes vont s'accentuer dans les prochaines années. Si le problème de la désertification médicale est évoqué depuis près de vingt ans, le plus important est encore à venir et les zones rurales ne seront pas les seules concernées. Par cet amendement du Sénat, la mobilisation de jeunes étudiants et professionnels dans les zones sous-dotées représente un levier d'action important pour résorber ou améliorer fortement-

L'accès aux soins ne saurait se réduire à la disponibilité des médecins. Nous savons que les ruptures de stock de médicaments se sont amplifiées au cours des dernières années : un Français sur quatre a déjà été confronté confronté à l'indisponibilité d'un médicament ou d'un vaccin. Sur l'initiative de Jean-Pierre Decool, le Sénat a mené une mission d'information à ce sujet l'été dernier. Madame la ministre, vous avez présenté la semaine dernière une feuille de route visant à mettre en oeuvre une partie des 30 propositions du

que de nombreuses pharmacies ne disposaient plus d'aucun corticoïde, médicament pourtant indispensable en premier recours pour de nombreuses maladies chez l'enfant et l'adulte. Il est toujours possible, bien sûr, d'adresser les patients aux urgences, mais celles-ci sont suffisamment encombrées. Toutes les actions d'amélioration sont donc absolument nécessaires, vont dans le bon sens et témoignent de notre volonté commune, madame la ministre, de répondre au principal défi sanitaire de la France, qui est de garantir l'accès aux soins dans tous les territoires.

territoriale et transversale, au travers des CPTS, les projets territoriaux de santé, les réseaux d'hôpitaux et les maisons de santé, qui devront fonctionner ensemble, en concertation avec les élus locaux et les ARS, pour trouver les bonnes réponses à chaque situation territoriale, à chaque bassin de vie, notamment en renforçant les services d'urgences et les Ehpad, avec une augmentation sensible des infirmiers et des aides-soignants. Cela est primordial pour la prise en charge des patients, en parallèle du nécessaire renforcement des effectifs de ces formations.

et de la médecine hospitalière, modernise le déroulement des études médicales et accompagne l'évolution des pratiques au travers de la numérisation de la santé, notamment avec le

à commencer par la levée progressive du, nous espérons une implication de l'hôpital et des facultés de médecine dans l'accès à la santé pour tous, en liaison avec les élus locaux et les CPTS, l'objectif étant

Traduction de la stratégie Ma Santé 2022, annoncée par le Président de la République le 18 septembre dernier, ce texte a pour ambition de transformer en profondeur notre système de santé pour assurer à chaque Français la qualité et la sécurité des soins. Réformer les études de médecine, notamment en supprimant le, réarticuler médecine de ville et hôpital, développer l'offre numérique, améliorer l'offre hospitalière de proximité, promouvoir les communautés professionnelles territoriales de santé : tels ont été les points centraux de nos discussions. deux assemblées n'avaient pas la même vision de ces enjeux, je me félicite de ce que les échanges en commission mixte paritaire aient abouti à un compromis, un texte équilibré qui reprend en particulier les avancées du Sénat, représentant des territoires, sur la lutte contre les déserts médicaux.

les critères de définition des besoins en professions médicales des territoires, discutés entre universités et ARS. Sur ces points, notre groupe restera attentif. Il le sera aussi sur les modalités modifiant l'accès au troisième cycle, et donc au choix de spécialité, avec le vote de la suppression de l'examen classant national actuel pour le remplacer par un dispositif qui, s'il visera à s'assurer du niveau de connaissances des étudiants, prendra également en compte les compétences cliniques acquises, les qualités humaines développées et l'ensemble du parcours des candidats. Mais si une réforme des études médicales a d'abord pour ambition de mieux former les étudiants, elle vise aussi à offrir aux territoires un meilleur accès aux soins. Comme vous l'avez dit vous-même, madame la ministre, cela « ne réglera pas le problème de la démographie médicale Aussi, je salue l'accord trouvé concernant la professionnalisation de la dernière année de l'internat de médecine. Proposé par les sénateurs soucieux d'assurer une prise en charge dans l'ensemble des territoires qu'ils défendent et représentent, cela prendra la forme d'un stage devant être effectué en ambulatoire, en priorité dans les zones sous-dotées, pendant six mois- contre un an dans la version initiale du dispositif sénatorial -, le tout encadré par un maître de stage. À À cet effet, les conditions pour devenir maître de stage ont été assouplies. Je salue tout autant la volonté de développer les CPTS, outil d'organisation donné aux professionnels du terrain, qui sont les mieux à même d'évaluer les besoins et d'élaborer les solutions de circuits de prise en charge de la population. Mes chers collègues, la notion et la prise en compte de la responsabilité populationnelle des professionnels de santé doivent être encouragées, car le médecin, l'infirmier mais aussi les aides-soignants et les kinésithérapeutes sont bel et bien des acteurs de santé publique. Je regrette toutefois que les avancées prévues par le Sénat n'aient pas été suivies en ce sens, notamment l'ambition de réaffirmer la notion d'infirmier référent, outil majeur dans le cadre d'une coordination des soins promue par les CPTS. Toujours dans l'objectif de simplifier la prise en charge coordonnée des personnes, le numérique- et les outils qu'il offre, notamment pour le suivi des patients -constitue un virage essentiel qu'il convient d'encourager, mais surtout de faciliter. Aussi, l'automaticité de l'ouverture du dossier médical partagé, ou d'un espace numérique de santé, l'ENS, permettra de déployer cet outil pour tous. Les acteurs de la santé pourront ainsi mieux prendre en charge, et de manière plus coordonnée, leurs patients. À ces fins, nos assemblées ont pu s'accorder sur la nécessité d'une offre de proximité de qualité. Les hôpitaux de proximité sont un des éléments forts du maillage territorial et de la vision d'un exercice coordonné de la médecine. La gradation des soins doit être vue non pas comme une médecine à deux vitesses, mais bien pour ce qu'elle est : une réorganisation d'un système à bout de souffle, comme l'ont montré les difficultés des services d'urgences qui s'amplifient, et une meilleure coordination ville-hôpital. Enfin, notre groupe se félicite des enrichissements du texte, qui bénéficieront aux territoires d'outre-mer, particulièrement en ce qui concerne l'autorisation d'exercer des praticiens à diplôme hors Union européenne. Le groupe s'est par ailleurs montré vigilant sur la question de Mayotte, où l'urgence sanitaire est on ne peut plus alarmante. Il le restera quant au financement de la future agence régionale de santé. Mes chers collègues, si cette nouvelle loi de structuration de l'offre de santé dans notre pays a pour objectif l'amélioration des conditions d'exercice de la médecine et d'accès aux soins, il faudra aussi penser dès la rentrée, avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, aux mécanismes de financement d'un tel projet qui devra s'inscrire dans la durée. Madame la ministre, vous avez avec beaucoup de sagesse montré la voie. Puisque M. Milon a cité Pascal et Mme Cohen Descartes, j'évoquerai quant à moi Confucius : quand le sage montre la lune du doigt, l'insensé regarde le doigt. Le groupe La République En Marche votera bien évidemment ce texte.

La question des difficultés de l'accès aux soins est devenue omniprésente dans la plupart des débats relatifs à la santé. En effet, la désertification médicale touche aujourd'hui l'ensemble de nos territoires. Si les centres urbains ont longtemps été épargnés par ce phénomène, on note aujourd'hui que même les grandes villes peinent à proposer une offre de soins satisfaisante pour leurs habitants.

que dans les organisations, certes nécessaires mais chronophages, et surtout prévues à des échelons qui n'incarnent en rien la proximité. Afin d'apporter une réponse concrète à ces difficultés, Corinne Imbert avait proposé à l'occasion de nos débats de transformer la dernière année du troisième cycle de médecine en une année de pratique ambulatoire en autonomie dans les zones sous-dotées. Loin de constituer une contrainte pour les internes en médecine, cette proposition avait pour objectif d'apporter une solution rapide pragmatique aux difficultés rencontrées dans nos territoires. Ce sont ainsi 3 500 étudiants, pour la seule médecine générale, qui auraient pu venir travailler en renfort aux côtés des médecins installés,

Deuxièmement, la durée d'un an aurait permis d'inscrire cet apprentissage professionnalisant en zones sous-dotées dans un temps long, optimisant ainsi l'éventualité d'une installation des internes dans ces territoires. enfin, la notion de pratique ambulatoire en autonomie est essentielle, car, contrairement à ce qui est d'usage dans un stage classique, le médecin n'aurait pas besoin d'être en permanence avec l'étudiant. L'effet direct serait d'augmenter le nombre de patients pris en charge. Cette proposition a d'ailleurs été reprise par d'autres groupes politiques du Sénat et votée par la quasi-totalité des sénateurs, ce qui illustre le caractère transpartisan et consensuel d'une telle mesure. Corinne Imbert remercie l'ensemble des sénateurs, qui, dans un esprit de défense de l'intérêt général et de l'intérêt de nos territoires, ont su mettre de côté leurs divergences idéologiques pour défendre collectivement une mesure de bon sens. bon sens. Non, le Sénat n'est pas tombé sur la tête ce jour-là ! Une nouvelle fois, il a fait honneur à sa réputation, à son esprit constructif et à la qualité de ses propositions. À force de discussions et d'échanges sur ce sujet, le Sénat et l'Assemblée nationale sont parvenus à un compromis, aux termes duquel chaque étudiant de dernière année de troisième cycle de médecine devra réaliser un stage de six six mois minimum dans un territoire sous-doté, en autonomie supervisée. Bien que cette mesure ne soit pas entièrement satisfaisante, elle est un début de réponse aux difficultés rencontrées par nos concitoyens. Dans les mois et années à venir, nous devrons être en mesure de proposer d'autres solutions innovantes afin de répondre à l'urgence rencontrée en matière d'accessibilité aux soins. Il n'y a pas une sénatrice ou un sénateur dans cet hémicycle qui n'ait été sollicité par un élu ou un administré sur cette thématique. La colère gronde, madame la ministre. Cela a déjà été dit. Entendez-la, avant que les solutions drastiques et caricaturales ne s'imposent d'elles-mêmes Le Sénat s'est également employé à renforcer la place des élus locaux dans le pilotage territorial de la santé. En effet, l'organisation territoriale de notre système de santé ne peut être pensée et exécutée par des structures souvent déconnectées des réalités du terrain. C'est pourquoi le Sénat a voté le renforcement des prérogatives du conseil de surveillance des établissements publics de santé, où siègent les représentants des collectivités territoriales. De la même manière, cinq maires seront désignés dans le cadre de la mise en oeuvre du projet régional de santé et de ses orientations, notamment sur l'accès aux soins et l'évolution de l'offre de santé. La Haute Assemblée est historiquement le lieu de représentation des territoires. Les sénateurs connaissent le caractère pluriel de notre pays et les spécificités de chaque département. Afin de tenir compte de cette diversité, le Sénat a voté des amendements à apporter de la souplesse aux dispositifs de structuration du système de santé. Les besoins spécifiques de chaque territoire seront donc pris en compte dans le cadre des projets territoriaux de santé. Malgré une commission mixte paritaire conclusive, que nous saluons, ce texte nous laisse un sentiment d'inachevé. En effet, de nombreuses mesures seront prises par ordonnance malgré la mise en garde des sénateurs. De la même manière, on peut regretter que ce texte ne réponde pas à la nécessité d'une restructuration de la gouvernance et du financement de notre système de santé. Lors des futurs textes de loi consacrés à la santé, vous pourrez compter, madame la ministre, sur la force de proposition que constitue le Sénat pour continuer à répondre à la problématique de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire français. Dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous aurons à coeur de discuter de certains dispositifs qui n'ont pu être adoptés lors de l'examen de ce texte en raison de leur impact financier. À titre d'exemple, l'exonération de cotisations sociales pour les jeunes médecins, dès lors qu'ils s'installent dans les trois ans suivant l'obtention de leur diplôme dans les zones déficitaires, pourra constituer une réponse au manque d'attractivité que connaît actuellement la médecine libérale. De la même manière, le financement des hôpitaux de proximité demeure encore incertain et il faudra apporter des précisions dans ce domaine. Ce débat fondamental aura également lieu, nous n'en doutons pas, lors de l'examen du projet

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous touchons ici à la dernière étape de l'examen d'un projet de loi qui focalisait tellement d'attentes de la part de nos territoires, marqués par la désertification médicale et par une crise de confiance sans précédent. Il aurait fallu aller plus loin, et vous le savez, madame la ministre, pour répondre à l'anxiété des élus locaux que nous rencontrons chaque semaine.

Cette concurrence malsaine entre territoires n'est pas à la hauteur du principe d'égal accès aux soins et laisse nombre d'élus locaux sans solution. La récurrence des grèves dans les urgences, en Sarthe et sur l'ensemble du territoire, démontre combien la situation est tendue. Comme l'a très bien exposé notre collègue Yves Daudigny, des avancées notables ont pu être obtenues grâce à l'apport du Sénat, notamment à l'article 2, obligeant les internes à effectuer, en dernière année de troisième cycle de médecine générale, un stage de six mois en ambulatoire prioritairement en zones sous-denses. Cette généralisation du Saspas, que nous avons proposée et qui a emporté notre non-opposition, pourrait avoir des effets concrets à court et moyen terme. À la différence de ladite « suppression » du, mesure de bon sens mais qui n'aura que peu d'effets directs et instantanés- cela a été également ce stage constitue l'une des solutions pour lutter contre le phénomène de désertification médicale. Les territoires attendent beaucoup de cette mesure emblématique de souche sénatoriale. Nous serons donc très vigilants quant à sa mise en place rapide par le Gouvernement. Autre point positif de cette loi, le développement de la télémédecine : il est évident que le télésoin peut apporter un service efficace et permettre de régler certaines situations délicates, notamment pour des publics incapables de se déplacer. Toutefois, je tiens à le rappeler fermement, la télémédecine ne peut se substituer à la présence physique d'un médecin. Sans parler des problématiques d'accès au numérique, lequel demeure un sujet dans nos territoires ruraux, le risque est évidemment de créer une médecine à deux vitesses, l'une présentielle pour les territoires attractifs, l'autre virtuelle pour les territoires délaissés et déjà impactés par la disparition excessive de services publics comme privés. À ce sujet, je ne me résous pas à l'abandon de l'article 13 A, qui introduisait un principe de médiation numérique en santé pour les usagers distants des nouvelles technologies, principe particulièrement pertinent en zone rurale et recommandé par le Défenseur des droits. Il n'est pas nécessaire, madame la ministre, de vous rappeler l'importance du maintien d'une offre de santé diversifiée au plus près des territoires. Je pense notamment à l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, qui peut être remis en cause par le simple départ à la retraite d'un gynécologue, comme ce fut le cas l'été dernier en Sarthe à l'hôpital du Bailleul. Alors que le sujet est extrêmement sensible et qu'une tribune de nos collègues députés vous appelle à inscrire dans notre Constitution ce droit à l'IVG afin de le protéger, il est étonnant de constater quelles sont les positions du Gouvernement et de la majorité à l'Assemblée Quand le Gouvernement exprime par votre voix, madame la ministre, un avis défavorable à l'extension des délais légaux d'accès à l'avortement, une mesure portée ici même avec pugnacité par notre collègue Laurence Rossignol, la majorité ne réintroduit pas le regretté article 27, qui tendait à demander à vos services un rapport sur l'accès effectif à l'IVG dans nos territoires. J'avais proposé à l'automne dernier de mettre sur pied un groupe de travail au sein de la commission des affaires sociales du Sénat ; en vain. C'est donc avec une réelle déception que je vois ce rapport abandonné, car il aurait permis de mettre en lumière les difficultés de beaucoup de femmes qui ne peuvent plus, en France, avoir accès à leur droit. Vous pouvez compter sur le groupe socialiste et républicain pour porter cette question de justice à chaque occasion jusqu'à ce que votre discours, volontariste, se concrétise enfin. Nous attendons plus de cohérence, madame la ministre Ainsi, loin de clore certaines questions, cette loi ouvre des débats dont nous serons amenés à reparler dans un avenir proche. Je pense notamment à la question des données et à celle du recueil du consentement des patients. Nous avons défendu le principe du consentement comme fondement de la licéité du traitement des données personnelles en santé, et donc de l'ouverture de l'espace numérique de santé, en lieu et place de l'ouverture automatique initialement prévue et portée par le groupe majoritaire. À l'heure où les croisements de données vont devenir exponentiels, il s'agit de replacer le patient au coeur du système et d'affirmer le principe de consentement libre et éclairé, qui n'en devient que plus fondamental alors que nous ne mesurons pas forcément les conséquences de l'utilisation des « applis » de santé et de bien-être. De manière identique, les modalités de création et de gestion du Health Data Hub, ou « plateforme des données de santé », ne sont pas suffisamment encadrées par le projet de loi. Nous aurons assurément l'occasion d'en reparler lors des débats à venir sur le projet de loi relatif à la

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du Gouvernement. Personne ne demande la parole ?

... L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement

au terme de plusieurs semaines d'échanges nourris avec nos collègues députés, je suis heureux de vous présenter un texte commun sur le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, biodiversité, issu des travaux de la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 25 juin dernier. Je rappelle que le texte initial visait trois objectifs principaux doter le monde de la biodiversité d'un opérateur public unique ; renforcer les attributions des agents dotés de prérogatives de police environnementale ; réformer l'organisation des activités de chasse en cohérence avec la création du nouvel établissement public. En première lecture, nous avions abordé ce projet de loi avec l'approche pragmatique et attentive aux besoins des territoires qui est la marque de notre assemblée, et l'avions significativement enrichi. Lors de la commission mixte paritaire, nous nous sommes montrés particulièrement soucieux de préserver l'équilibre délicat que le Sénat avait ainsi construit. Le texte de compromis qui en résulte conserve l'essentiel de nos apports, et nous pouvons nous en féliciter.

président du groupe d'études « Chasse et pêche », de leur engagement à mes côtés et de leur contribution au texte que nous examinons aujourd'hui. Sur notre initiative, des améliorations importantes ont été apportées à la gouvernance du nouvel établissement public succédant à l'Agence l'ONCFS, afin de garantir une représentation plus équilibrée des différentes parties prenantes. En particulier, nous avons introduit une représentation des organisations professionnelles agricoles et forestières, fixé un quantum minimal pour la représentation des acteurs de la chasse et de la pêche et posé le principe d'une présence minoritaire de l'État en nombre de représentants, équilibrée par la création d'un commissaire du Gouvernement doté d'un droit de veto. de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, ne saurait conduire à une dégradation des ressources des agences de l'eau. C'est un ajout très important au regard des inquiétudes que nous avons tous sur l'avenir de la politique de l'eau. À ce sujet, nous ferons preuve d'une vigilance toute particulière, vous le savez, madame la secrétaire d'État, sur la traduction budgétaire de la création de l'OFB à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2020. En matière de police de l'environnement, notre travail s'est inscrit pleinement en continuité de l'approche retenue par l'Assemblée nationale, en apportant des précisions aux attributions des inspecteurs de l'environnement. Nous avons eu le même souci de renforcer les pouvoirs des inspecteurs et de ne pas disperser les compétences de police. Une autre priorité du Sénat a été de consacrer et d'amplifier la contribution du monde de la chasse à la protection de la biodiversité. Nous avons ainsi précisé le système de financement d'actions en faveur de la biodiversité par les fédérations des chasseurs et inscrit dans la loi l'engagement pris par l'État de soutenir ces actions à hauteur de 10 euros par permis de chasser. Le dispositif équilibré auquel nous sommes parvenus permettra de conforter les nombreuses actions menées au quotidien par les fédérations de chasseurs pour une gestion durable de la biodiversité. Néanmoins, Néanmoins, il nous appartiendra de rester très vigilants sur l'utilisation de ces fonds et sur une solidarité qui devra s'exprimer entre les fédérations départementales. Madame la secrétaire d'État, j'ai eu l'occasion de vous le dire, nous comptons aussi sur votre vigilance en ce domaine. Le Sénat a également adopté plusieurs dispositions pour renforcer la lutte contre les dégâts de grand gibier, qui constituent un véritable fléau dans de nombreux territoires, en particulier pour pour les agriculteurs et les propriétaires forestiers. Je pense notamment à l'encadrement des pratiques de nourrissage et du transport des sangliers vivants, ainsi qu'au renforcement des pouvoirs du préfet à l'égard des plans de chasse en cas d'augmentation importante des dégâts. Nous avons en outre permis aux fédérations régionales des chasseurs d'être gestionnaires de réserves naturelles. Sur ce sujet, je tiens toutefois à préciser que, à titre personnel, je ne suis pas favorable à la mise en place d'une participation à l'hectare, tel que cela a été décidé. Il m'aurait paru plus judicieux de porter le permis national à 250 euros par exemple, ce qui représentait une large économie par rapport à son coût précédent, voisin de 400 euros. Je pense, je suis même persuadé, que cela aurait posé moins de problèmes financiers et d'organisation pour indemniser les dégâts de grand gibier. Parallèlement, c'est également au Sénat qu'ont été adoptées deux mesures importantes en matière d'encadrement des activités cynégétiques, prévoyant une harmonisation réglementaire des règles de sécurité et créant un régime de rétention ou de suspension du permis de chasser en cas de comportement particulièrement dangereux. Cela témoigne d'une approche très exigeante et responsable de la chasse, en vue d'assurer la sécurité de tous et de permettre une coexistence encadrée et sereine des différentes activités dans nos territoires. Enfin, nous avons adopté plusieurs dispositions concrètes en faveur d'une meilleure protection du patrimoine naturel. Je pense notamment à des ajouts précisant les critères de reconnaissance des zones humides, élargissant le périmètre des aires marines protégées et introduisant dans la loi une définition de la géodiversité. L'ensemble de ces évolutions ont été apportées en tenant pleinement compte du travail effectué par l'Assemblée nationale. Les dispositions que nous avons adoptées s'ajoutent à celles qui par nos collègues députés, de façon cohérente et constructive, avec le même souci de proposer une réforme durable en matière de biodiversité. Sur le fondement de ces travaux, nous avons oeuvré activement avec Mme Barbara Pompili, rapporteure de l'Assemblée nationale, pour trouver un accord. Je tiens à saluer le travail que nous avons accompli ensemble en commission mixte paritaire, ainsi que l'implication de notre président de commission, Hervé Maurey, qui est retenu aujourd'hui par une réunion de l'Union interparlementaire. Un point particulier a suscité des débats nourris jusqu'au dernier moment : l'introduction en première lecture au Sénat, sur l'initiative de notre collègue Jean-Noël Cardoux, d'un délit d'entrave aux activités de chasse, sujet d'actualité Je rappelle que, sur cette question, la volonté du Sénat était d'affirmer clairement l'impérieuse nécessité d'assurer le respect par tous des activités de chasse et de pêche dûment autorisées. Un certain nombre d'exactions insupportables envers les chasseurs et les pêcheurs, des menaces et des dégradations de leur équipement, sont régulièrement constatées. Cela participe plus globalement d'une remise en cause violente de certaines activités légales par une minorité radicale. L'objectif de l'introduction d'un délit d'entrave était de sanctionner spécifiquement ces comportements, avec des peines proportionnées à la gravité des faits. Bien que nous estimions cette disposition parfaitement fondée,

après que vous vous êtes engagée, madame la secrétaire d'État, conjointement avec le ministre chargé des relations avec le Parlement, à examiner avec attention la proposition de loi déposée par notre collège Jean-Noël Cardoux, traitant la question du délit d'entrave de façon plus transversale. Sous réserve de la décision de la conférence des présidents qui se réunira demain, ce texte devrait être inscrit à l'ordre du jour du Sénat en octobre. Nous serons particulièrement attentifs à ce que l'engagement pris par le Gouvernement se concrétise par une inscription rapide du texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Au-delà de cette question, nous avons élaboré- vous l'aurez compris, mes chers collègues -un texte de compromis, conservant les nombreux ajouts du Sénat que j'ai mentionnés à l'instant, aussi bien

concessions, lorsque les textes des deux assemblées différaient significativement sur certains points, mais je pense que nous pouvons collectivement être fiers de l'importante contribution du Sénat au texte que nous avons à examiner aujourd'hui et que je vous invite à adopter. La parole

et qui a fait l'objet- vous l'avez rappelé -d'une proposition de loi, portée par le sénateur Cardoux. Vous avez annoncé la possibilité d'une inscription rapide de ce texte à l'ordre du jour du Sénat ; le Gouvernement s'est engagé à faciliter son examen rapide à l'Assemblée nationale pour que ce sujet puisse être traité de façon transversale.

Cet établissement réunira 2 700 agents aux compétences complémentaires sur l'eau et la biodiversité, marine et terrestre, rassemblés dans un établissement unique pour une action plus forte, mieux coordonnée, sur tous les territoires. Il sera au service du ministère. Nous allons retravailler ses liens avec les services déconcentrés et les autres opérateurs pour la mise en oeuvre de ses politiques en matière d'eau et de biodiversité. L'office sera particulièrement mobilisé

nous avons accru les pouvoirs des inspecteurs de l'environnement, qui pourront, sous contrôle du procureur de la République, conduire leurs enquêtes de la constatation de l'infraction au renvoi du prévenu devant le tribunal, sans avoir à se dessaisir au profit d'un officier de police judiciaire généraliste. bénéficieront d'un cadre de collaboration amélioré avec les autres services de police. Les peines sont renforcées pour les délits d'atteinte aux espèces et habitats protégés et pour le délit d'exercice illégal aggravé de la chasse.

nationale ont adopté ces mesures en commission mixte paritaire -des obligations minimales de sécurité homogènes au niveau national, un dispositif de rétention et de suspension du permis de chasser en cas de manquement grave à une règle de sécurité et une obligation de formation pour les accompagnateurs de jeunes chasseurs. Nous avons aussi progressé sur la question de la maîtrise des dégâts de gibier, en suivant les recommandations de la mission du député Alain Perea et du sénateur Jean-Noël Cardoux : interdiction du nourrissage des sangliers et restriction des lâchers dans les enclos, ce qui permettra également de lutter contre l'engrillagement notamment observé en Sologne. La loi incite financièrement les chasseurs à mieux réguler le grand gibier, en faisant davantage sur les territoires de chasse où les dégâts sont les plus importants.

Pour ces espèces, la déclaration des prélèvements par chaque chasseur sera obligatoire auprès des fédérations de chasseurs et de l'OFB. La loi instaure une éco-contribution afin que les fédérations de chasseurs financent chaque année, à hauteur de 5 euros par chasseur, des actions concrètes en faveur de la biodiversité, comme la plantation de haies, la restauration de milieux forestiers et de milieux humides, l'entretien d'habitats favorables à la biodiversité. Des crédits publics cofinanceront ces actions à hauteur de 10 euros pour 5 euros de contribution par chasseur.

Après relecture attentive du texte issu de la CMP, nous avons noté quatre erreurs ou oublis de coordination. Le Gouvernement a donc déposé quatre amendements pour les corriger, lesquels seront examinés à l'issue de cette discussion générale, et qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale mardi dernier.

Sur le premier point, je souhaite vous assurer que la totalité du besoin de financement nécessaire pour faire face à la baisse du permis de chasse sera assurée par des voies budgétaires, ce qui permettra de ne pas effectuer de prélèvements sur les agences de l'eau. Cette inquiétude avait été exprimée à de nombreuses reprises pendant les débats : je suis donc maintenant en mesure de vous affirmer que les agences de l'eau ne connaîtront aucune perte de recettes associée à la création du nouvel établissement et à sa budgétisation. sa budgétisation. Comme dans n'importe quel rapprochement d'établissements, des questions légitimes sont posées par les personnels et leurs syndicats, que j'ai d'ailleurs reçus la semaine dernière. Nous avons avancé sur la possibilité d'effectuer une requalification

Je m'en félicite, car rien n'était acquis au vu des différends notoires exprimés dans les nombreux amendements déposés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Finalement, les mesures les plus clivantes ont été dans leur grande majorité supprimées ou aménagées par la commission mixte paritaire. Et bien qu'ayant défendu certaines d'entre elles, je ne vais pas m'opposer au texte que nous avons à voter. Je tiens à souligner la véritable volonté de compromis des rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que du Gouvernement, mais aussi l'excellent travail effectué en amont par le groupe d'études « Chasse et pêche ». Ce projet de loi corrige une anomalie qui n'avait pu être réglée lors de l'adoption de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, portée par Ségolène Royal, car le projet d'intégration de l'ONCFS dans l'Agence française de biodiversité était alors combattu par l'ensemble du monde de la chasse, dont je faisais partie. Aujourd'hui, tout est différent. L'accord passé entre le Président de la République et le président de la Fédération nationale des chasseurs, la fixation du prix du permis national à 200 euros et la contribution des chasseurs, couplée à celle de l'État, au nouveau fonds pour la protection de la biodiversité, a permis à cette fusion d'être désormais acceptée par la majorité des parties prenantes. Cette opération s'inscrit en effet dans la continuité de la stratégie nationale pour la biodiversité. Mon collègue Jean-Michel Houllegatte l'affirmait ici, lors de la discussion générale de la première lecture du texte, « nous sommes convaincus qu'il existe entre le monde de la chasse et la protection de la nature une convergence des objectifs et une complémentarité justifiant la fusion de ces deux établissements »,

Tout au long de l'examen du texte, je me plais à le souligner, les sénateurs du groupe socialiste n'ont cessé de défendre une vision équilibrée du futur établissement. Attentifs à ce que ce dernier soit le plus fédérateur possible, nous nous sommes attachés à préserver ses missions essentielles de protection de l'environnement, mais surtout à prendre en compte les attentes des différentes parties prenantes. nous avons défendu un certain nombre d'amendements en ce sens. Nous avons notamment milité pour que le monde agricole et forestier figure expressément au sein du conseil d'administration de l'Office. l'inscription dans le texte de la contribution de 10 euros de l'État, en contrepartie de celle de 5 euros des chasseurs, dans le cadre de la création du futur fonds pour la protection de la biodiversité, a également été soutenue et portée par le groupe socialiste. Ma conviction profonde est que la gestion de ce fonds, confiée à la Fédération nationale des chasseurs, permettra à celle-ci de mener à bien la lourde tâche de protection et de reconquête de la biodiversité, tout en sachant prendre en compte, je l'espère, les attentes et les souhaits des fédérations départementales des chasseurs. Enfin, le groupe socialiste a fait adopter l'affectation à titre gratuit à l'OFB de biens mobiliers dont, à l'occasion d'une décision de justice, la propriété avait été transférée à l'État, ainsi que des mesures permettant de renforcer la lutte contre les dégâts causés par le grand gibier. Lors de l'examen du texte, j'ai été particulièrement attentif à ce dernier point. En effet, le département dont je suis élu, la Dordogne, est directement touché par ces dégâts, le plus souvent occasionnés par des sangliers. Je me réjouis d'ailleurs du travail mené

Toutes ces mesures serviront, j'en suis convaincu, à rendre plus fort et efficient le nouvel Office. Toutefois, il me paraît nécessaire, mes chers collègues, d'appeler votre attention sur un certain nombre de points.

Vous le savez, je suis un défenseur de la chasse populaire. Dans mon département, la Dordogne, j'ai été sollicité par de nombreux chasseurs qui n'étaient pas convaincus par la baisse du prix du permis de chasse national couplée à la disparition du permis bi-départemental. Ces chasseurs doivent aujourd'hui s'acquitter du permis national pour chasser dans le département voisin, et cela représente une hausse tarifaire discriminante pour les chasseurs les plus modestes. Cette question doit être étudiée le plus rapidement possible par la Fédération nationale des chasseurs, comme elle s'y est engagée ; j'attends une réponse très rapide de sa part. Il nous Il nous faudra également rester attentifs, mes chers collègues, au respect de toutes les parties prenantes au sein du conseil d'administration de l'Office. Le droit de veto accordé au Gouvernement en contrepartie d'une participation minoritaire ne doit pas mener à des abus qui seraient préjudiciables au bon fonctionnement de l'OFB.

susceptibles d'être chassés », introduite par le Sénat, ait été supprimée, au motif qu'elle relevait d'une loi de finances. Ce dispositif ayant vocation à devenir la principale source de financement des fédérations départementales des chasseurs, en remplacement du timbre national grand gibier, il sera nécessaire

et nous serons, une fois encore, très attentifs à ce que l'État tienne ses engagements. Je conclus, mes chers collègues, en saluant de nouveau la qualité du travail parlementaire lors de l'examen de ce projet celui-ci ne soit pas parfait et qu'il reste des zones à éclaircir, notamment en matière de financement, le groupe socialiste votera majoritairement pour l'adoption de ce texte. La parole

Je ne peux donc que me réjouir du succès de cette commission mixte paritaire, et je salue le travail des rapporteurs et des présidents de commission. Ce succès grave ainsi dans la loi cette fusion nécessaire, et le groupe du RDSE votera très majoritairement en faveur des conclusions de la de loi permet en effet de doter notre pays d'un outil plus puissant pour tenter de faire face à cet enjeu majeur, la préservation de notre patrimoine naturel, et pour participer à la définition d'une stratégie efficace visant à stopper la perte de la biodiversité, une menace pour l'avenir même de nos sociétés. Il convient maintenant que ce nouvel office s'investisse résolument dans la définition de cette stratégie, avec comme priorité la préservation des écosystèmes. Cela nécessite de trouver enfin les leviers permettant d'en finir avec les pollutions chimiques et le gaspillage insensé de terres agricoles et naturelles. L'enjeu de l'artificialisation des terres, qui fragilise notre futur et notre autonomie alimentaire, sera d'ailleurs inclus dans une proposition de résolution que mes collègues Françoise Laborde et Joël Labbé défendront en octobre prochain, dans le cadre d'une niche du groupe du RDSE. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir, mais ce débat est déjà l'occasion d'exprimer l'attente, que je crois assez partagée sur les travées du Sénat, d'une loi efficace contre l'artificialisation des sols. Cet exemple me semble en effet assez symptomatique du fait que chasseurs et écologistes ont plus d'intérêts communs qu'ils ne l'affichent. J'avoue d'ailleurs avoir été quelque peu déçu de la teneur du débat que nous avons eu au Sénat, au cours duquel beaucoup d'amendements adoptés par la majorité sénatoriale

tolérer demain des chasses non sélectives. L'Espagne a déjà été condamnée par l'Union européenne sur ce fondement et des recours européens ont aussi été déposés par des associations françaises. Plus généralement, certaines pratiques, largement rejetées par la population, jouent contre l'image de la chasse ; elles réduisent les vocations alors que nous avons besoin de chasseurs pour réguler certaines populations de gibier, en particulier de sangliers. Je ne désespère pas, chers collègues, que nous ayons un jour un débat serein et sans tabou sur cette question de l'image de la chasse, laquelle se considère trop comme une citadelle assiégée, se battant pied à pied sur les listes d'espèces chassables ou les dates de chasse, alors que l'enjeu est d'abord la synergie entre

Deux sujets seront d'ailleurs l'occasion de l'approfondir. D'abord, la contribution de 10 euros par chasseur cotisant, que l'État s'apprête à créer au bénéfice de l'action « biodiversité » de la Fédération nationale de chasse, fait aujourd'hui, vous le savez, grincer bien des dents chez les associations de protection de l'environnement. Il appartiendra donc aux chasseurs de faire mentir les procès d'intention sur l'utilisation de ce que d'aucuns dénomment « le chèque fusion la gestion adaptative des espèces constituera un autre test. Le principe est intéressant, et, effectivement, cette approche par espèce donne satisfaction dans d'autres pays. sur ce point aussi, c'est bien l'application qui en sera faite concrètement qui montrera l'existence, ou non, de convergences entre chasseurs et protecteurs de la nature. Soit il s'agit de limiter la pression de chasse sur des espèces fragiles, à la population en déclin, comme la tourterelle des bois, le courlis cendré ou la barge à queue noire,

qui dit gestion adaptative dit suivi scientifique. Le CEGA, le Comité d'experts sur la gestion adaptative, a préconisé un moratoire

justifié. Je profite de cette intervention pour souligner que, sans moyens, les politiques de reconquête de la biodiversité ne peuvent être couronnées de succès. Ainsi, les ponctions régulières sur les recettes des agences de l'eau ne sont plus acceptables, tant le budget de ces organismes est nécessaire aux politiques de restauration des milieux humides.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, chers collègues, les membres de la commission mixte paritaire sont parvenus à un accord sur une version commune du projet de loi créant l'Office français de la biodiversité ; c'est une heureuse nouvelle. Idée ancienne, longtemps controversée, cette fusion de deux grands établissements publics- l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage concourent, chacun avec sa culture et ses moyens, à la préservation de l'environnement permettra, en mutualisant les ressources et les compétences, de renforcer l'efficacité des actions menées sur tout le territoire français,

Cette fusion répond à de nombreux objectifs. Parmi ceux-ci, j'en note trois : replacer les enjeux des politiques environnementales à un échelon territorial- cela doit intéresser les sénateurs -, faire converger l'action des politiques de l'eau et de la biodiversité- quand on voit les problèmes que connaît notre pays dans le domaine de l'eau, il n'est pas inintéressant de s'en préoccuper -et renforcer les pouvoirs de police de l'environnement. Cela permet d'achever le travail de fusion des opérateurs de la biodiversité

Je me félicite du maintien de plusieurs dispositions que j'avais proposées en faveur d'une meilleure protection du patrimoine naturel. Je pense notamment aux ajouts précisant les critères de reconnaissance des zones humides et élargissant le périmètre des aires marines protégées ; cela témoigne indéniablement de la reconnaissance de l'importance des zones humides dans la préservation de la biodiversité. Je me réjouis également du renforcement des pouvoirs de la police environnementale. Les diverses mesures relatives à ces pouvoirs devraient améliorer les conditions de travail des agents, concrètement, sur le terrain et dans leur vie de tous les jours. Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, enrayer l'effondrement de la biodiversité est plus que jamais capital ; ces deux notions vont évidemment de pair, et l'ajout de la mention du changement climatique à l'article 1 est essentiel. Le changement climatique contribue directement aux considérables pertes de biodiversité, mais il constitue également un facteur d'aggravation de certaines causes indirectes.

La protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique doivent donc être deux combats menés de front par la France et par l'ensemble de la communauté internationale. Comme pour le climat, les solutions

Nous devrons veiller à ce que l'OFB ait bien les moyens humains et financiers d'agir efficacement et concrètement. Nous avons en effet le talent formidable de construire des outils magnifiques, mais parfois, par une bizarrerie propre

Le travail en bonne intelligence avec toutes les parties intéressées- agriculteurs, acteurs économiques, chasseurs, organismes privés et publics, ONG, scientifiques -devra se poursuivre, car il sera primordial pour le bon fonctionnement de ce nouvel office et pour le succès de ses missions.

à le souligner, l'économie générale de l'accord conclu entre le Président de la République et la Fédération nationale des chasseurs a été respectée. Je citerai, en vrac, le permis à 200 euros, la gestion adaptative, l'éco-contribution, la police de l'environnement ; tous ces dossiers, que la FNC avait portés, ont été préservés et maintenus dans le texte. En outre,

avons un sentiment d'inachevé sur certains dossiers. Je ne reviendrai pas plus longuement sur ce fameux délit d'entrave, qui a créé beaucoup de crispations et

par la rapporteure de l'Assemblée nationale, de la sanctuarisation des chasses traditionnelles et de la prise en compte de la notion de chasse durable pour la mise en oeuvre de la gestion adaptative.

auraient beaucoup d'argent et peut-être peu de projets, et, inversement, les petites fédérations, ayant peu d'argent parce qu'elles comptent peu de chasseurs, ne pourraient pas financer leurs projets. Je suis de ceux qui croient que l'argent de l'eau doit aller à l'eau

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

À contre-courant des attentes de nos concitoyens, certains auraient bien voulu transformer ce texte important pour la biodiversité en texte pour la chasse et pour les chasseurs. Néanmoins, c'est avec soulagement que nous accueillons finalement ce compromis, proche du texte de l'Assemblée Le projet de loi, qui vise à renforcer les moyens de l'action publique pour défendre la biodiversité, n'a pas été, au bout du compte, trop dévoyé. C'est un soulagement, car certaines dispositions votées au Sénat étaient de nature à aggraver l'effondrement en cours de la biodiversité. Je pense notamment à l'autorisation de techniques d'un autre temps, comme la chasse à la glu, ou à l'extension de la chasse aux oiseaux migrateurs, proposées alors même que la France a perdu près du tiers de ses oiseaux depuis le début du siècle. Je peux rassurer mes amis chasseurs : ils seront toujours autorisés à chasser une vingtaine d'espèces d'oiseaux menacés et pourront même chasser deux nouvelles espèces. C'est également un immense soulagement de voir disparaître l'odieux délit d'entrave à la chasse, qui remettait en cause qui remettait en cause l'accès pour tous à la nature et ravivait des clivages inutiles entre les différents usagers. Les trop nombreux accidents de chasse ayant coûté la vie à des promeneurs nous rappellent qu'une réflexion devra être menée, pour garantir à chacun un accès, en toute sécurité, à l'espace naturel, qui constitue notre patrimoine commun. Ces scories retirées, nous pouvons nous féliciter du renforcement des prérogatives des inspecteurs de l'environnement, des nouvelles dispositions permettant de mieux protéger la biodiversité ultramarine ou de celles permettant de lutter contre la biopiraterie. Nous saluons la création d'un établissement unique doté de moyens mutualisés, bien qu'insuffisants, pour agir au service de la reconquête de la biodiversité, souhaitée par toutes les associations de protection de l'environnement depuis le Grenelle.

alors même que le nouvel office manque de moyens financiers, que l'on ponctionne encore le budget des agences de l'eau pour le financer, que la suppression des postes d'inspecteurs de l'environnement se poursuit et que l'on déplore des trous dans la raquette en termes de maillage territorial. Nous espérons que le prochain budget actera le début des subsides promis à l'époque par Nicolas Hulot, à savoir 600 millions d'euros supplémentaires pour le plan Biodiversité. Vous n'avez pas jugé opportun, madame la secrétaire d'État, de les inscrire dans le dernier projet de loi de finances, préférant créer ce nouvel office avec un déficit structurel de près de 40 millions d'euros. d'euros. Nous vous demandons de rassurer la représentation nationale sur ce point. Vous venez de le confirmer, il n'y aura pas de nouveaux prélèvements sur les agences de l'eau, ce dont je me félicite. La sanctuarisation du budget de l'OFB est indispensable. Ponctionner les agences, c'est limiter les investissements en matière d'eau potable et d'assainissement, donc agir moins en faveur de la biodiversité. Ce serait un comble, au moment où l'on demande aux intercommunalités de prendre la compétence eau et assainissement et où les besoins d'investissements sont croissants, alors même que les Assises de l'eau mettent en lumière d'importants besoins liés aux conséquences des changements climatiques sur l'état et la répartition des masses d'eau ! Comme je l'évoquais en première lecture, le Gouvernement est devenu spécialiste en « plomberie administrative » : on réorganise, tout en espérant améliorer l'action publique à moyens constants, voire pire, avec moins de moyens. On doit vous reconnaître un certain talent dans la gestion de la pénurie. Néanmoins, quelle que soit l'efficacité opérationnelle du nouvel office, il ne pourra pas grand-chose sans moyens, et notamment sans moyens humains. Les syndicats de personnel dénoncent un plan social : la suppression de 127 postes, soit 5 % des effectifs. Triste incohérence ! Allez-vous stopper l'hémorragie humaine que connaît votre ministère ? serait une nécessité pour déployer correctement l'Office dans les territoires. Le débat parlementaire n'aura malheureusement pas permis de lever cette inquiétude, pourtant soulevée dès la première lecture par la rapporteure à l'Assemblée nationale. Dans de nombreux départements, les effectifs planchers de l'office ne sont pas atteints. La présence des agents sur le terrain est pourtant la raison d'être d'une telle administration, qui ne pourra pas préserver la biodiversité depuis des bureaux parisiens. Il faudra des agents sur le terrain, notamment pour déployer le plan Loup, qui est censé soutenir et accompagner le pastoralisme, améliorer les connaissances et expérimenter de nouvelles méthodes, indemniser les éleveurs et réguler les populations de loups

Ayant présenté un certain nombre d'amendements en faveur d'une meilleure gouvernance, partagée entre tous les usagers et les professionnels des espaces naturels- j'entends par là les chasseurs, mais aussi les forestiers et les agriculteurs -, je regrette, pour l'efficacité et l'équilibre de l'OFB, que certaines dispositions aient finalement été retirées de ce texte. tenir à l'écart de l'Office français de la biodiversité et de la gestion des plans de chasse les propriétaires agricoles ou forestiers, acteurs, selon moi, légitimes des territoires ruraux, ne me semble pas une posture souhaitable et durable. l'intérêt d'ignorer des problématiques de multiusages bien réels, qui ne feront que s'exacerber ? Je pense notamment à l'amendement qui visait à prévoir la compatibilité entre les plans de chasse et les plans d'aménagement des forêts publiques, au regard des dégâts croissants de gibier sur des massifs forestiers affaiblis- on le voit aujourd'hui -par des déficits croissants et de plus en plus vulnérables aux attaques parasitaires. Quel est l'intérêt de refuser une gestion durable et partagée, responsabilisant l'ensemble des acteurs des territoires ? Ainsi, en matière de gouvernance, le seuil minimum de 10 % des membres du conseil d'administration représentant les organisations professionnelles agricoles et forestières a été supprimé. Il demeure toutefois possible de déléguer des compétences du conseil d'administration à des commissions spécialisées. Nous comptons donc sur la sagesse des décisionnaires de l'OFB, qui les conduira, je l'espère, à s'emparer de ces options d'équilibre qui figurent encore dans le texte, pour une gouvernance plus légitime et, donc, plus durable au service de la biodiversité. Il en est ainsi de la levée de l'obligation de constituer une réserve dans une ACCA pour le grand gibier gibier ; de l'avis de la Commission régionale de la forêt et du bois pour fixer le nombre du grand gibier soumis au plan de chasse ; des pouvoirs renforcés du préfet pour lutter contre les dégâts du grand gibier

ce que nous attendons tous dans les plus brefs délais, vu les tensions sociétales qui se manifestent aujourd'hui pour la chasse, comme pour d'autres activités pourtant régulièrement autorisées. a également supprimé l'extension de la contribution à l'hectare aux territoires « susceptibles d'être chassés », ce qui risque, malheureusement, de créer des comportements d'aubaine. Elle a rétabli la rédaction de l'Assemblée nationale sur l'encadrement du droit d'opposition à l'intégration d'un terrain dans une ACCA, une association communale de chasse agréée, en contradiction, je l'avais dit, avec une décision du Conseil d'État d'octobre 2018, fondée sur la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En matière de financement, elle a tout de même confirmé le souhait du Sénat, en sanctuarisant les ressources des agences de l'eau, vous l'avez dit, madame la secrétaire d'État. Elle a précisé le schéma de financement des actions en faveur de la biodiversité, en retenant le principe d'une contribution des fédérations départementales à un fonds géré par la Fédération nationale et dont l'utilisation sera déterminée par convention. Enfin, elle a maintenu l'engagement de l'État à soutenir les efforts des fédérations à hauteur de 10 euros par permis de chasser validé dans l'année, en visant explicitement la réalisation des actions de protection ou de reconquête de la biodiversité. Le texte final apporte donc un certain nombre d'avancées, sans écarter pour autant l'épée de Damoclès qui pèse désormais dangereusement sur la biodiversité en forêt, à savoir l'augmentation massive de dégâts de gibier dans un contexte, je l'ai dit, de vulnérabilité sans précédent des forêts, alors que le Gouvernement, dans le cadre du programme national de la forêt et du bois, incite à exploiter plus.

Prince. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'adoption du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité par la commission mixte paritaire du 25 juin dernier est une très bonne nouvelle. La création de ce nouvel office permettra de renforcer et de rendre plus effective la lutte pour la sauvegarde, sur notre territoire, de la biodiversité, qui est aujourd'hui menacée. On ne peut donc que se féliciter de l'accord trouvé par les représentants des deux chambres, tant le sujet est important et l'attente de nos concitoyens, forte. La fondation de l'OFB permettra une répartition plus homogène des équipes sur le terrain. Les représentants des chasseurs et pêcheurs entreront dans la gouvernance de l'établissement. Ils pourront ainsi s'impliquer mieux dans la réponse aux problématiques liées à la protection de la biodiversité. Les moyens de police de l'environnement pourront être mutualisés pour une meilleure efficacité. La gestion adaptative des espèces, processus permettant de redéfinir cycliquement la gestion d'une espèce selon l'état de sa population, assurera une meilleure gestion de la biodiversité. À ce sujet, la commission a su trouver une position équilibrée quant aux obligations de transmission de données incombant aux chasseurs. Le délit d'entrave à la chasse, qui avait été voté au Sénat, a finalement été retiré du texte. Son adoption aurait permis de sanctionner les individus empêchant ou gênant les chasseurs. Néanmoins, le Gouvernement s'est engagé à ce que la proposition de loi de notre collègue Cardoux, qui vise à sanctionner plus largement l'entrave aux activités légales, soit examinée devant les deux chambres. L'idée d'apporter une réponse pénale adéquate à cet inquiétant phénomène n'est donc pas abandonnée et fera l'objet d'une discussion au Parlement dans le cadre d'un véhicule législatif dédié. Autre point positif : la discussion de ce texte a été l'occasion d'alerter sur la question de l'engrillagement. La pose sauvage de clôtures porte atteinte aux écosystèmes des milieux naturels. En Sologne, on compterait déjà 3 600 kilomètres de clôtures. Il est nécessaire que les élus se saisissent de cette question, qui peut être réglée au niveau des collectivités lors de l'élaboration des documents d'urbanisme. En outre, si elle a abandonné l'extension des missions des fédérations départementales des chasseurs à la répression du braconnage, la commission a en revanche renforcé les pouvoirs du préfet dans le cadre de la lutte contre les dégâts de grand gibier. Sur le plan financier, les recettes destinées aux actions en faveur de la protection et de la restauration de la biodiversité sont définies avec une plus grande précision : il s'agit d'une éco-contribution de 5 euros par permis de chasser et de 10 euros par l'État La commission mixte paritaire a également maintenu avec raison la sanctuarisation des ressources des agences de l'eau votée au Sénat. Malgré les engagements pris, la question des ressources de l'établissement demeure posée. Je veux croire toutefois que le Gouvernement fournira à l'Office les moyens de mener correctement les missions qui lui ont été confiées. Vous venez d'ailleurs de nous le confirmer, madame la secrétaire Les défis qui attentent l'OFB sont importants. En mai dernier, un rapport rédigé par un comité d'experts de l'ONU s'alarmait de la disparition de la biodiversité, menacée par des facteurs multiples, dont la déforestation, une utilisation trop intensive des ressources naturelles, la pollution ou encore les espèces exotiques invasives. Il est temps que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour enrayer ce phénomène d'extinction de la biodiversité, qui menace notre patrimoine commun, mais aussi nos économies et notre alimentation. Le groupe Union Centriste votera en majorité pour ce texte. La parole est à Mme Anne Chain-Larché. Monsieur

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, aboutir à un accord en CMP pour le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement n'était pas gagné d'avance, tant s'en faut. Je tiens à remercier mes collègues Jean-Claude Luche et Jean-Noël Cardoux pour le travail qu'ils ont accompli. Le texte que nous examinons contient en effet de nombreuses dispositions introduites par le Sénat, ce dont je me félicite. Tout d'abord, la CMP a conservé nos principales propositions en matière de gouvernance de l'Office français de la biodiversité. Cet établissement issu de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage était très attendu. Le Sénat avait été particulièrement attentif à la place des chasseurs au sein de ce nouvel établissement. Les chasseurs sont des acteurs incontournables en matière de développement et de protection de la biodiversité. Il nous avait donc semblé normal qu'ils bénéficient d'une représentation minimale au sein du conseil d'administration. Le texte prévoit ainsi d'octroyer 10 % des sièges aux représentants des chasseurs et des pêcheurs. L'État, quant à lui, ne disposera pas de la majorité au sein du nouvel établissement, mais uniquement d'un droit de veto. Il devra savoir convaincre ses partenaires et rechercher le consensus. Ce système fonctionnait parfaitement à l'ONCFS, et je ne doute pas qu'il en sera de même au sein du nouvel établissement. Autre disposition à laquelle nous tenions : l'inscription dans la loi de l'engagement pris par l'État de contribuer à hauteur de 10 euros par permis de chasser aux actions réalisées par les fédérations de chasseurs en faveur de la biodiversité. Cet engagement de l'État permettra ainsi d'amplifier les projets que mènent déjà les chasseurs. Par ailleurs, un dispositif de péréquation entre la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales dotées d'un faible nombre d'adhérents sera également mis en oeuvre. Cela devrait rassurer les fédérations départementales qui s'étaient inquiétées de l'impact d'un permis de chasser à 200 euros et des conséquences d'une taxe à l'hectare rendue obligatoire. Autre sujet d'importance : la sécurité à la chasse. Chaque accident est un accident de trop. Le Sénat avait voté des dispositions permettant d'harmoniser les pratiques. Elles sont maintenues dans le texte, ce dont nous nous félicitons. La CMP a également sanctuarisé les ACCA, ce qui est une bonne chose, car celles-ci contribuent au développement du gibier et de la biodiversité, en favorisant le regroupement de terrains morcelés de petite taille. Leur rôle n'est plus à démontrer. Elles sont la garantie d'une chasse populaire qu'il faut absolument maintenir. Mais aboutir à un accord de la CMP suppose des concessions de part et d'autre. C'est savoir renoncer à des dispositifs auxquels nous tenions tout particulièrement. Le Sénat a pris ses responsabilités. ce qui concerne la dénomination du nouvel établissement, issu de la fusion entre l'ONCFS et l'AFB, puisque le mot « chasse » disparaît. Souhaitons que ce ne soit pas de mauvais augure pour le monde cynégétique. Tel est également le cas du délit d'entrave à la chasse. C'est une question extrêmement importante pour les chasseurs et qui nous concerne tous. Notre collègue Jean-Noël Cardoux a déposé une proposition de loi permettant de réprimer l'ensemble des entraves à l'exercice des libertés. Le Gouvernement a estimé que ce texte constituait un véhicule plus adapté pour aborder la question du délit d'entrave à la chasse. Je souhaite que le Sénat s'en saisisse dès la rentrée et qu'il soit examiné par les députés dans des délais rapides, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement.

Vous avez pris, madame la secrétaire d'État, des engagements devant la Haute Assemblée. Nous vous avons entendue. Nous comptons sur vous pour trouver des solutions de financement pérennes pour l'OFB, tout en permettant aux agences de l'eau de réaliser leurs investissements en matière d'eau potable et d'assainissement. nous serons particulièrement attentifs aux décisions qui seront prises lors du prochain budget. En attendant, nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la création de ce grand établissement public qu'est l'Office français de la biodiversité témoigne d'une volonté collective de préserver la biodiversité. C'est une dynamique qu'on ne peut que saluer.

deux établissements publics : l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'Agence française pour la biodiversité, issue elle-même d'une fusion de quatre établissements réalisée voilà moins de deux ans.

remercie de cet engagement auquel le monde rural est sensible. La violation du droit de propriété par des activistes vegans, sur des terrains de chasse, mais aussi sur des exploitations agricoles, est de plus en plus fréquente. Cette situation inacceptable est réellement préoccupante. Il faut donc agir pour préserver

L'année 2020 sera une année importante pour la biodiversité, puisque le Congrès mondial de la nature se tiendra à Marseille. Par ailleurs, une conférence

les effectifs, je vous redis l'attention toute particulière que je porte au personnel, afin de trouver la bonne organisation, pour parvenir à quelques gains de productivité sur les fonctions support, au moment du rapprochement, en particulier au plan national, et maintenir les agents au plus près du terrain. Pour les agents de développement, vous avez raison, nous devons trouver la bonne articulation- nous continuerons à la chercher. De même, nous n'avons pas épuisé la totalité des sujets forêt et ACCA, mais nous continuerons à y travailler. C'est donc un beau texte, équilibré, qui porte réforme de la chasse ; un texte qui permettra d'avancer sur les sujets liés

de la biodiversité. Contre toute attente, un accord a été trouvé. Le texte de la CMP permet une représentation plus équilibrée des différentes parties prenantes. Madame la secrétaire d'État, vous avez précisé que le conseil d'administration comprendrait entre 30 et 40 membres. C'est un progrès par rapport au projet initial. J'avais d'ailleurs proposé par amendement que la loi fixe ce nombre à 30. Autre évolution : l'État ne sera plus majoritaire mais décidera avec tous les acteurs concernés. Ces avancées vont dans le sens d'une pluralité nécessaire au bon fonctionnement de l'Office. Concernant les outre-mer, nous partions de loin ! Je rappelle que le texte initial ne comportait aucune référence aux territoires aux territoires ultramarins. Un non-sens, quand on sait que 80 % de la biodiversité se trouve dans les collectivités d'outre-mer et que la France abrite, avec ces mêmes territoires ultramarins, 10 % des espèces connues au niveau mondial. La Nouvelle-Calédonie à elle seule est considérée comme le deuxième de la planète en matière de biodiversité, et 75 % des récifs français sont calédoniens. Eu égard à l'immense richesse de la biodiversité ultramarine, il était inconcevable que ce projet de loi fasse l'impasse sur les outre-mer. Grâce à l'action des parlementaires, nos territoires ont trouvé une place dans ce dispositif la représentation des Ultramarins et des bassins écosystémiques sera assurée dans le conseil d'administration. Mais, j'y insiste, une fois que la nouvelle structure sera mise en place, elle devra assurer la participation effective des outre-mer. Je partage l'inquiétude de notre collègue Michel Magras sur l'absence de référence à un comité d'orientation dédié à la biodiversité ultramarine. Il faut à tout prix maintenir un espace de dialogue au coeur de l'OFB. Le futur office ne doit pas être une simple fusion de deux opérateurs. Il doit représenter toutes les parties, être le lieu de débats et porter une ambition nouvelle, à la hauteur de l'immense enjeu qu'est la biodiversité.

explication de vote. J'avais en première lecture voté contre le texte tel qu'il était issu du Sénat. Je reconnais bien volontiers que le texte de la commission mixte paritaire revient sur un certain nombre de dispositions que

leurs représentants coalisent l'ensemble des intérêts des différentes chasses, parce que, le plus souvent, ce n'est pas de toutes que l'on parle. Dans mon département, chaque année, pendant les périodes de chasse, il y a des incidents graves entre les riverains de la forêt et les veneurs, puisque les grands animaux se réfugient dans les jardins, dans les centres-villes à présent, et, à chaque fois, la population prend la défense des grands animaux

en épingle. Vous dites que les veneurs squattent les forêts : ils sont, dans ces forêts domaniales, adjudicataires et parfaitement en règle ; ils ont le droit de chasser. Depuis ces incidents, la société de vénerie et la fédération nationale des chasseurs ont élaboré une charte

Le scrutin est ouvert.

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018

on n'a laissé que quelques jours au Sénat pour auditionner le ministre, examiner les 43 articles additionnels introduits à l'Assemblée nationale et rédiger les amendements de la commission.

Il y a en effet urgence. Partout, les signaux passent au rouge. Le vivant dans son ensemble s'érode. Comme nous le savons tous, la planète se réchauffe, et, avec elle, les conditions de notre pérennité risquent de s'éteindre également. L'examen du projet de loi Énergie-climat s'inscrit dans ce contexte particulier. Durant le grand débat, les Français ont réaffirmé leurs exigences et leurs attentes. Le scrutin européen a confirmé la préoccupation, chaque matin plus grande, de Voilà quelques jours encore, un épisode caniculaire exceptionnel nous rappelait que le dérèglement climatique peut bousculer nos économies, notre lien social, nos cultures, notre santé. Aujourd'hui, nous vivons un épisode de sécheresse ; soixante et Il faut regarder la réalité en face. L'heure est à l'action. Un seul sujet doit importer : répondre à l'urgence, relever le défi de la transition écologique. En un sens, ce qui se joue, c'est bien l'avenir de la planète.

Pour répondre à une telle urgence, le Président de la République a souhaité que l'ambition écologique soit au coeur de l'acte II du quinquennat. Le Premier ministre l'a précisé dans son discours de politique générale au mois de juin : les mois à venir devront être ceux de l'accélération écologique. Aller encore plus loin, c'est notre ambition. Elle s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale du Gouvernement et du ministère de la transition écologique et solidaire. Depuis le début du quinquennat, le Gouvernement a mis fin à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures. Il a mis en place des aides au bénéfice des Français, notamment des plus modestes, pour changer leurs manières de se déplacer, de se chauffer, de se loger.

d'énergies- nous commençons par le principe de sobriété et de réduction de la consommation -, un développement massif des énergies renouvelables et la réduction de la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Nous avons également défendu à l'échelon européen et international le renforcement des normes environnementales favorables au climat et à la biodiversité. Plus récemment, nous avons travaillé avec toutes les parties prenantes dans les Assises de l'eau pour engager en deux phases des actions concrètes pour renouveler les réseaux, protéger les captages et économiser la ressource en eau. Le projet de loi que vous examinez aujourd'hui amplifie et prolonge cette ambition écologique. Il comporte quatre objectifs principaux, que je souhaite rappeler ici. Le premier est de permettre la publication et l'adoption de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la mise en oeuvre de notre stratégie énergétique pour les dix années à venir. Le deuxième objectif est de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, rehausser nos objectifs climatiques et adapter notre gouvernance pour les atteindre. Pour ce faire, à l'article 1, nous fixons l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. En termes de méthode, il s'agit de diviser les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six par rapport à 1990 ; c'est donc plus ambitieux que le texte actuel. Nous diminuerons encore davantage notre consommation énergétique primaire d'énergies fossiles, en passant avec cette loi de moins 30 %, qui est la base législative actuelle, à moins 40 % d'ici à 2030. Nous avons également souhaité mettre en place une instance d'expertise scientifique indépendante. Le Haut Conseil pour le climat, créé à l'article 2 de la loi, sera chargé d'émettre des avis et recommandations sur l'ensemble des politiques publiques et sur leur conformité avec notre trajectoire climatique ambitieuse. Comme vous le savez, cette instance a commencé ses travaux et nous incite à aller plus loin et à mieux intégrer les enjeux écologiques dans toutes nos politiques publiques. Le troisième objectif de ce texte est de nous donner les moyens d'assurer la fermeture des centrales à charbon en accompagnant les territoires et les salariés concernés. Le Président de la République en a pris l'engagement. C'est un choix fort pour le climat. Ces quatre centrales émettent près de 10 millions de tonnes de CO2 par an, soit à peu près l'équivalent de 4 millions de véhicules thermiques. L'article 3 du texte donne au Gouvernement l'assise juridique nécessaire pour procéder à la fermeture effective des centrales, en permettant à l'autorité administrative de plafonner leur durée de fonctionnement. Depuis dix mois, nous mettons tout en place pour nous donner les moyens juridiques, humains et territoriaux pour réussir cette mutation industrielle et accompagner les territoires et les salariés concernés. Notre objectif est de signer les projets de territoire sur les quatre territoires touchés avec les élus, les parties prenantes et les acteurs économiques d'ici à la fin de l'année 2019. Enfin, le quatrième objectif est de régler des problèmes trop longtemps restés en suspens. En matière d'autorité environnementale, l'insécurité juridique qui demeurait jusqu'alors favorisait les contentieux et fragilisait les petits projets d'énergies renouvelables, notamment solaires. L'article 4 doit permettre de sécuriser le cadre juridique de l'évaluation environnementale, afin de faciliter la concrétisation des projets en revenant au système en vigueur jusqu'alors. Des dispositions ont été adoptées à l'Assemblée nationale pour accélérer plus encore le développement des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. Je m'en réjouis, pour la transition énergétique, pour nos territoires et pour les entreprises qui en bénéficieront. Sur les tarifs de l'électricité, le Gouvernement a pris des engagements forts devant les Français : geler les hausses en hiver et augmenter le montant du chèque énergie pour atténuer les effets des augmentations. Gouvernement, nous ne pouvons pas nous résoudre à être spectateurs d'un mode de calcul invariable. C'est pourquoi le projet de loi doit permettre de stabiliser les prix en relevant le plafond de l'Arenh à 150 térawattheures, ce qui permettra aux consommateurs français de profiter de la stabilité des prix du parc nucléaire. Nous avons aussi fait procéder à une saisine rectificative du Conseil d'État pour que les éléments de la loi Pacte concernant les tarifs régulés du gaz et de l'électricité puissent être adoptés dans le cadre de ce projet de loi.

Je sais que les parlementaires aspirent à être pleinement associés à la politique énergétique. C'est légitime, et j'y souscris. Le principe d'une loi de programmation quinquennale pour le climat répond à cette attente. Cette loi vous sera présentée à la prochaine échéance de la PPE, en 2023. Tous les cinq ans, le Parlement aura les moyens de s'assurer de la réussite de la transition énergétique et d'en fixer les prochaines étapes. C'est une évolution significative par rapport à la loi de 2015. En bref, le texte qui vous est présenté aujourd'hui sera l'occasion de renforcer l'implication et le travail du Parlement, afin que celui-ci joue pleinement son rôle dans la transition écologique. Parmi les mesures supplémentaires que les députés ont souhaité introduire, je pense à la question essentielle de la rénovation des passoires thermiques sont une aberration écologique et représentent évidemment un coût pour nos concitoyens. C'est pourquoi, pour agir sans pénaliser les propriétaires, le texte a prévu trois phases : incitation, obligation, contrainte. Cette dernière phase sera définie lors de la programmation quinquennale de l'énergie en 2023. La convention citoyenne pour le climat pourra évidemment être associée à ces réflexions et proposer des mesures pour en accélérer le mouvement. Dans la première période, l'incitation, avec Julien Denormandie, nous retravaillerons à la simplification des aides, à l'amélioration des dispositifs d'accompagnement des particuliers, à l'amélioration de l'accompagnement des professionnels, à la gestion des copropriétés, pour en faire en sorte que le système soit le plus fluide, le plus opérationnel et le plus efficace possible. possible. Les amendements que le Gouvernement défendra au cours des débats visent principalement à préciser des éléments techniques, notamment sur la rénovation, sur les garanties d'origines et, plus largement, sur les tarifs du gaz et de l'électricité. De plus, nous avons souhaité soutenir l'hydrogène décarboné, produit à partir de l'électrolyse de l'eau, suite à de nombreuses demandes, pour profiter pleinement du mix électrique français. Nous souhaitons véritablement garantir l'efficacité de l'autorité environnementale à travers son organisation. C'est un impératif pour pouvoir atteindre nos objectifs en matière d'énergies renouvelables. Enfin, le Gouvernement doit conserver la possibilité de relever le plafond de l'Arenh. Nous en avons pris l'engagement devant les Français. Avant le débat en séance, le texte qui nous rassemble aujourd'hui a pu bénéficier de l'expertise des sénatrices et des sénateurs en commission. Je comprends que les délais ont été très brefs. Je voudrais saluer l'investissement de tous ceux qui y ont travaillé jusqu'à présent. Je vous remercie Je vous remercie aussi d'avoir été constructifs, car nous avons l'occasion de trouver ensemble des terrains d'entente et de construire une vision et un plan d'action véritablement durables. Je crois pouvoir le dire, le travail a été riche, qu'il s'agisse de compléter la définition de la neutralité carbone, d'intégrer l'aspect social dans le plan stratégique d'EDF ou d'apporter des améliorations le contrat expérimental pour les solutions électriques renouvelables innovantes. De nombreuses autres précisions et simplifications soulignent la connaissance fine de nombre d'entre vous sur ces sujets. vous sur ces sujets. Mesdames, messieurs les sénateurs, je crois qu'il revient naturellement au législateur de fixer les orientations de long terme de la politique énergétique et climatique et au Gouvernement de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour les réaliser. Ce texte répond à la nécessité que nous agissions et que chacun prenne ses responsabilités. Déjà enrichi par le débat parlementaire, il constitue une étape décisive dans la transition écologique. Je forme le voeu que les débats qui s'ouvrent aujourd'hui soient constructifs, ce sera le cas. Je serai à vos côtés dans ce débat. Nous ne devons avoir qu'une seule bataille, une seule exigence : relever le défi de la transition écologique. C'est

malgré l'inflation du nombre de ses articles, la « petite loi énergie » l'est encore, sans conteste, par son manque de vision stratégique à long terme. C'est sûr ! Le Gouvernement a dit s'inscrire dans le prolongement de la loi de transition énergétique de 2015, mais cela n'empêchait ni l'ambition ni la volonté d'embrasser tous les grands sujets de la politique énergétique. Or nombre de ces sujets sont absents du texte. Je pense en particulier aux enjeux de compétitivité de nos entreprises, car l'énergie est un poste important de leur budget, pour les industries intensives en énergie, bien sûr, mais pour toutes les entreprises en général. Je pense aussi à la manière dont nous pourrions mieux gérer nos formidables ressources de biomasse, qu'elles soient agricoles ou forestières, et mieux exploiter le potentiel de capture du carbone par nos sols et nos forêts. Je pense encore aux énergies renouvelables, au biogaz, à l'éolien, au solaire, à l'hydroélectricité, grande ou petite, ou à la géothermie, que le champ très restreint du texte déposé ne nous a permis que d'effleurer,

mais encore faut-il savoir comment on y parvient. En la matière, le texte ne comportait qu'une seule mesure concrète- la fermeture des quatre dernières centrales à charbon d'ici à 2022 -, qui n'y suffira pas. Comme si l'essentiel était renvoyé à la convention citoyenne pour le climat, et si le Gouvernement comptait se défausser sur des citoyens tirés au sort ... En s'inscrivant dans la mécanique de la loi de 2015, ce texte organise aussi le dessaisissement du Parlement on nous demande d'entériner dans la loi des évolutions décidées à l'avance, dans un projet de décret. En inversant ainsi la hiérarchie des normes, c'est un vrai problème de démocratie que l'on pose. Fort heureusement, grâce aux initiatives combinées de l'Assemblée nationale et de notre commission, c'est la dernière fois que nous vivons une telle situation : pour la prochaine PPE, c'est bien le Parlement qui fixera le cap et les priorités d'action, et ce sont la PPE et la stratégie bas-carbone qui seront chargées de les décliner ! Nous allons encore plus loin, en corrigeant une autre anomalie démocratique : celle qui fait que, aujourd'hui, c'est par simple décret qu'est fixé le volume des CEE, qui représentent pourtant plus de 3 milliards d'euros par an prélevés sur les consommateurs, soit 3 % à 4 % de leurs dépenses d'énergie. En 2023, c'est la loi qui fixera ce volume, sur la base d'une évaluation du gisement faite par l'Ademe. En matière de nucléaire, la loi a au moins le mérite de reconnaître que la date de 2025 était non seulement irréaliste, mais surtout contre-productive sur le plan du climat, puisqu'il aurait fallu faire appel à des moyens thermiques supplémentaires pour assurer notre approvisionnement. Mais, désormais, c'est la question du nouveau nucléaire qu'on laisse en suspens, alors que le GIEC juge lui-même que le nucléaire fait partie des solutions pour limiter le réchauffement climatique. Dans le cadre contraint fixé par les articles du texte initial, notre commission a cherché à promouvoir sa vision d'une bonne politique énergétique. Pour donner de la visibilité aux filières dans lesquelles la France a encore une carte industrielle à jouer, nous avons fixé des objectifs ambitieux, ambitieux, mais réalistes : atteindre au moins 27 gigawatts de capacités hydroélectriques installées en 2028 ; augmenter les capacités d'éolien en mer d'au moins un gigawatt par an d'ici à 2024, pour traduire dans la loi l'annonce faite par le Premier ministre dans son discours de politique générale cibler 8 % de biogaz en 2028 pour respecter l'objectif des 10 % fixé par la loi en 2030, alors que ce n'est pas le chemin que prend la PPE, ce qui est quand même un comble Sur le soutien au biogaz, j'entends bien les considérations budgétaires ; nous y sommes très attentifs, car c'est toujours le consommateur d'énergie qui paie à la fin. Mais j'observe qu'on consacre 7 milliards à 8 pour l'électricité renouvelable, parfois pour des filières qui sont matures ou en passe de l'être, et que, dans le même temps, on hésite à mettre les quelques centaines de millions nécessaires au démarrage d'une filière non intermittente, riche en emplois localisés et porteuse de nombreuses externalités positives. Certes, comme en toute chose, il faut éviter les excès et s'assurer de la disponibilité de la ressource à l'échelle locale. Pour accompagner nos industries françaises et européennes, ce sont aussi nos dispositifs de soutien qu'il faut revoir. Notre commission a voulu poser un principe : la prise en compte dans tous les mécanismes d'aides publiques du bilan carbone des projets. On veut mesurer notre empreinte carbone dans tous les secteurs. Il n'y a pas de raison que les énergies renouvelables fassent exception. Au contraire ! C'est leur objet même de décarboner notre énergie. Ce sera bon pour le climat et pour nos entreprises. Le droit européen ne s'y oppose pas, pourvu que ce bilan carbone soit analysé de manière transparente et non discriminatoire. Pour encourager l'essor des énergies renouvelables, la commission a aussi consolidé ou ajouté plusieurs dispositifs, que ce soit pour simplifier encore les augmentations de puissance des installations hydroélectriques concédées, sans remise en concurrence ; faciliter le déploiement de centrales photovoltaïques sur les sites dégradés en zone littorale ; ou concilier le développement du solaire au sol aux abords des routes avec la préservation des surfaces agricoles. Pour ne pas déstabiliser la filière du biogaz, nous avons aussi reporté de dix-huit mois la réforme des garanties d'origine et prévu un accès privilégié des collectivités à ces garanties pour préserver le lien avec les territoires. Sur ce point, je vous proposerai d'aller encore plus loin en séance. En matière de rénovation énergétique des logements, la commission a souhaité tourner la page de la mise sous séquestre, qui avait un temps été imaginée à l'Assemblée Elle a réaffirmé la primauté de l'incitation, de l'information et de l'accompagnement sur la sanction. Non seulement la contrainte touche aussi les propriétaires occupants ou bailleurs aux revenus modestes, mais elle se révèle souvent contre-productive, notamment parce qu'elle sort un grand nombre de logements du marché. Nous avons donc renforcé l'information des locataires et des acheteurs, en ajoutant notamment le montant des dépenses théoriques dans le DPE, tout en rendant les dispositifs plus progressifs, avec un report à 2024 du conditionnement de la révision des loyers en zone tendue à l'atteinte d'une certaine performance énergétique. La commission a aussi cherché à mieux accompagner les salariés concernés par la fermeture des centrales à charbon, ainsi que les consommateurs dans le cadre de la fin totale ou partielle des tarifs réglementés. Pour les premiers, nous avons réaffirmé le rôle de l'État dans la mise en place des mesures de reclassement et dit qu'il devra être tenu compte, quand ce sera possible, du statut des salariés. Pour les consommateurs, nous avons réintroduit le principe, déjà voté par le Sénat dans la loi Pacte, d'un prix de référence indicatif du gaz, qui sera calculé par la CRE et qui pourra servir de point de repère. sur l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'Arenh, la solution proposée par le Gouvernement répond à l'évidence à un enjeu de court terme, celui d'éviter la hausse des tarifs en cas d'atteinte du plafond. Elle n'exonère pas d'une réforme globale d'un système qui est aujourd'hui à bout de souffle. Sur ce point comme sur la réorganisation envisagée d'EDF, nous serons vigilants, je pense, sur toutes les travées, pour qu'un élément fort de notre patrimoine commun ne soit pas remis en cause. En attendant, et même s'il s'agit d'une solution transitoire, on ne peut pas passer par pertes et profits la juste rémunération du parc historique. Pour concilier cet objectif avec celui, tout aussi légitime, de la stabilité des prix, la commission a lié le relèvement du plafond à la révision du prix et a mentionné explicitement la prise en compte de l'inflation, puisque le prix n'a pas évolué depuis 2012. On nous dit que la Commission européenne n'acceptera jamais la révision du prix. Si tel était le cas, pourquoi le Gouvernement fait-il croire que cette révision pourrait avoir lieu ? Très bien ! Par ailleurs, si l'on explique à la Commission que ce sera la révision du plafond et du prix sinon rien, nous serons en position de force pour négocier, sachant que la simple prise en compte de l'inflation est une revendication raisonnable et, me semble-t-il, parfaitement audible par Bruxelles. Au total, mes chers collègues, même si le texte n'a pas l'ambition que nous aurions souhaitée, la commission l'a adopté après l'avoir amendé dans le sens que je viens de vous présenter : de la visibilité et du soutien pour nos filières de l'industrie verte,

pour lequel la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a reçu une délégation au fond de la commission des affaires économiques de neuf articles, notamment l'article 2, sur le Haut Conseil pour le climat, et l'article 4 sur l'autorité environnementale. C'est une chance que deux commissions permanentes se soient penchées sur le berceau de votre politique énergétique. En effet, avec une seule petite semaine, le Sénat n'a pas disposé, le regrette, du délai suffisant pour examiner en profondeur ce texte, surtout avec quarante-trois articles additionnels.

Pour autant, elle ne saurait nous conduire à voter dans une hâte excessive un texte dont l'objet premier serait l'obtention d'un satisfecit médiatique. Il est facile d'annoncer de grands objectifs, encore faut-il être capable de transformer ces ambitions en réalité concrète. À cet égard, je déplore le manque d'une dimension territoriale dans ce texte, s'agissant, en particulier, du volet du soutien financier aux actions des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre,

S'agissant de la réforme de l'autorité environnementale, vous prétendez clarifier la situation à la suite de la décision du Conseil d'État d'annuler l'attribution au préfet de région de la compétence d'autorité environnementale responsable de l'évaluation de la qualité des études d'impacts réalisées. Loin de sécuriser les porteurs de projets, cette réforme risque pourtant de conduire à une multiplication des recours, compte tenu de l'absence d'autonomie de l'instance chargée d'examiner au cas par cas les projets par rapport à celle qui est compétente pour les autoriser. Notre commission a donc souhaité sécuriser le dispositif retenu au regard du droit européen, en limitant les situations potentielles de conflit d'intérêts. Enfin, je tiens à insister sur le manque d'anticipation du Gouvernement sur tous les plans.

La priorité absolue est d'assurer la production d'une énergie décarbonée. Il est encore plus risqué de prendre de telles décisions sans prévoir des dispositions spécifiques en faveur des milliers de salariés concernés par ces fermetures. Nous avons donc souhaité, avec mon collègue Daniel Gremillet, renforcer les mesures d'accompagnement de ces salariés. Madame la secrétaire d'État, je ne crois pas être hors sujet en évoquant la sempiternelle question du mix énergétique. Ce projet de loi et la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont le décret se fait attendre, s'appuient sur des hypothèses qui ne semblent pas gravées dans le marbre. Dès son introduction, la PPE considère qu'« en 2050, la consommation d'électricité décarbonée pourrait atteindre entre 580 et 610

ce projet de loi valide des options technologiques qui pourraient nous conduire dans une impasse énergétique à moyen terme. Nous n'avons pourtant qu'un horizon : décarboner notre production électrique. Je le dis sans enthousiasme, les leviers ne sont pas inépuisables.

réponse. Je déplore que ce texte, voté si rapidement, nous prive d'un véritable débat de fond sur notre politique énergétique. Je forme le voeu que, à l'avenir, nous puissions débattre au Parlement de cette question si essentielle de manière moins expéditive.

le projet de loi relatif à l'énergie et au climat qui nous est soumis aujourd'hui a d'abord pour fonction de permettre de publier la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Comme la PPE ne prévoit pas de baisse significative de la part du nucléaire dans les prochaines années, elle entrait en effet en contradiction avec la loi en vigueur, laquelle imposait la réduction rapide

signe de l'incapacité française à s'engager résolument dans la transition énergétique et comme une traduction de notre difficulté à concevoir la sortie en bon ordre de notre dévotion au dieu atome, dans lequel nous avons investi bien au-delà du raisonnable, comme l'histoire est en train de le démontrer. En ce sens, je souhaite saluer les apports de la majorité sénatoriale et du rapporteur Daniel Gremillet, qui a intégré dans le texte la nouvelle ambition française dans le domaine des énergies renouvelables et notamment de l'éolien offshore ou du gaz renouvelable.

de le souligner. Il s'agit d'une loi sur l'énergie et le climat. Est-il nécessaire de souligner que la question climatique est aujourd'hui un sujet central ? Tout ou presque a été dit sur le sujet. Ce que nous ne disons peut-être pas assez, c'est que l'enjeu de la réduction des émissions de CO2 françaises est une brique essentielle de la mobilisation mondiale.

Comment voulez-vous réussir à embarquer les autres pays vers le respect de l'accord de Paris si vos émissions augmentent, comme ce fut le cas entre 2015 et 2017 ? Je souligne ce point, car un des arguments dilatoires les plus entendus,

Malheureusement, sur ces points, le Sénat n'a guère renforcé le projet de loi. Le débat à l'Assemblée nationale n'avait déjà pas brillé par le volontarisme à propos de la rénovation énergétique des bâtiments anciens et les trous dans la raquette étaient nombreux.

Or, aujourd'hui, les poids lourds étrangers se soustraient de plus en plus aux péages autoroutiers en empruntant les routes nationales et départementales. Ce report de trafic cause d'importantes difficultés, notamment dans les départements frontaliers tels que la Moselle. C'est à partir de ce constat, à la fois national et local, que je souhaite aujourd'hui défendre le retour au système de l'écotaxe sur les poids lourds. En effet, le projet d'écotaxe, qui a été malheureusement abandonné en novembre 2016, constituait un instrument pertinent de politique des transports et une réponse aux enjeux climatiques, écologiques et sanitaires actuels. Il s'agit d'appliquer deux principes simples : celui de l'utilisateur-payeur, selon lequel les transporteurs routiers s'acquitteraient d'un droit d'usage, comme c'est le cas pour le rail,

Certes, la ministre des transports a annoncé le 9 juillet que le remboursement partiel du gazole dont bénéficie ce secteur sera réduit de 2 centimes par litre. Toutefois, cette mesure est insuffisante. De plus, elle est injuste, puisque, dans les faits, les poids lourds étrangers y échapperont en faisant le plein de carburant au Luxembourg ou en Espagne, ce qui leur permettra de traverser la France sans y acheter une goutte de gazole. Compte tenu des défis environnementaux que nous devons relever, il nous faut être plus ambitieux et développer des instruments plus stratégiques pour mettre réellement en oeuvre la transition énergétique dans nos territoires.

ce qui ne permettra peut-être pas d'y apporter la contribution qu'il aurait méritée. En outre, ce projet de loi aurait pu être plus ambitieux, car les enjeux sont très importants et urgents. Je voudrais remercier nos rapporteurs et nos administrateurs, qui, malgré des conditions difficiles, ont fait un travail remarquable. travail remarquable. Ce texte confirme l'objectif d'une réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production d'électricité et le report de son échéance à 2035 au lieu de 2025. Cette proposition me paraît réaliste, car l'objectif initial était inatteignable. Il prévoit la fermeture des centrales à énergies fossiles, notamment de celles qui fonctionnent au charbon, en 2022. C'est une mesure positive, car, si la part du charbon dans la production d'électricité n'est que de 1,8 %, sa part dans les émissions de gaz à effet de serre est de 35 %.

prévu pour encadrer la reconversion des salariés de ces centrales, qui vont perdre leur emploi- ce sera le cas aussi pour les sous-traitants -, et l'accompagnement des territoires concernés. Un autre sujet essentiel traité est la politique de rénovation énergétique des bâtiments. Le secteur du bâtiment représente en effet 45 % de l'énergie finale consommée en France et 27 % des émissions de gaz à effet de serre. Rénover le parc permettrait d'endiguer ce problème. La solution est de mettre en place et de financer un vaste plan de rénovation énergétique des logements. Ces travaux doivent être de grande ampleur et ne pas concerner uniquement le remplacement des fenêtres ou le changement des chaudières. C'est à ce prix que nous pourrons atteindre la neutralité carbone en 2050. Concernant la question des passoires énergétiques dans les logements mis en location,

J'aimerais évoquer rapidement la filière éolienne, puisque la programmation pluriannuelle de l'énergie reprend l'objectif de développement des énergies renouvelables et renforce les trajectoires établies, en prévoyant ainsi, pour l'éolien terrestre, l'installation de 9 à 10 gigawatts par période de cinq ans. Si les objectifs d'installation d'éoliennes et de capacité solaire- 50 gigawatts à l'horizon de 2028 - doivent compenser la diminution de la production nucléaire, force est toutefois de constater que la gestion des énergies renouvelables devient très complexe lorsque leur taux de pénétration dépasse 30 % du mix énergétique.

du maintien d'une ambition importante de développement de l'éolien offshore, qui constitue un signal fort en faveur du développement de capacités industrielles nationales dans une filière en cours de structuration au niveau mondial.

le Sénat est contraint d'examiner le projet de loi Énergie-climat dans un temps très court, trop court. Cette petite loi de huit articles est devenue, sous la double action de l'Assemblée nationale et du Gouvernement, une petite loi de cinquante-six Nous regrettons vivement le calendrier imposé sur ce texte, madame la secrétaire d'État, qui ne permet pas l'examen de ses dispositions dans de bonnes conditions. Nous saluons, d'ailleurs, la proposition de redonner au Parlement son pouvoir de définition des objectifs stratégiques

du groupe Les Indépendants sont, par exemple, convaincus que le mix français doit être composé d'un bouquet d'énergies dont les sources différentes assureront autant la complémentarité que la fiabilité de l'approvisionnement énergétique. Parvenir à ce bouquet implique une diversité d'installations de production d'énergie. À ce titre, nos convictions portent sur trois points : nous encourageons toutes les énergies renouvelables, notamment l'énergie hydroélectrique, en laquelle nous croyons, en conciliation avec les utilisateurs des territoires nous plaidons pour une plus grande autonomie des territoires et de leurs élus, qui sont les mieux à même de résoudre les difficultés locales ; enfin, nous souhaitons anticiper dès aujourd'hui la mise à niveau, puis le démantèlement des installations. L'évolution rapide des technologies nous oblige à penser les sujets majeurs que sont les friches et la dépollution. Les enjeux sont technologiques, écologiques, mais aussi sociaux. Les emplois détruits par la fermeture de sites de production sont enfin sérieusement

Les Français nous ont rappelé avec force que l'écologie du quotidien, sur laquelle le Gouvernement souhaite faire reposer l'axe II du quinquennat, devra être ambitieuse et concrète. La lutte contre les passoires thermiques doit, par exemple, être intensifiée, parce que nous ne pouvons accepter que près de la moitié des logements privés en location soient notés F ou G. Rappelons-le, en la matière, l'énergie la plus écologique demeure celle qui n'est consommée. Un certain Président de la République disait il y a plus de quinze ans : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Les jeunes générations nous invitent aujourd'hui à garder les yeux bien ouverts et braqués dans la bonne direction.

nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le projet de loi relatif à l'énergie et au climat, dont l'objectif principal est d'accélérer la transition énergétique de notre société. Il s'agit bien d'une accélération, mes chers collègues, tant, depuis 2017, le Gouvernement oeuvre quotidiennement à cet objectif.

développement de solutions de mobilité plus propres, avec le renforcement de la prime à la conversion, le forfait mobilité durable, les dispositions sur les zones à faible émission, les objectifs de renouvellement des flottes, autant de mesures comprises dans le projet de loi Mobilités, dont vous venez, hélas, mes chers collègues, de faire échouer la commission mixte paritaire. Par ailleurs, le Gouvernement a engagé, dès juin 2017, la révision de la stratégie nationale bas-carbone, visant un objectif de long terme : la neutralité carbone dès 2050. Il s'est enfin attelé à la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie. outil de pilotage de la politique énergétique de la France a été créé par la loi de 2015 de transition énergétique pour la croissance verte. L'ensemble des piliers de la politique énergétique et des énergies y sont traités. Alors, mes chers collègues, vous pardonnerez mon étonnement, quand j'entends que cette « petite loi » serait dépourvue de « vision stratégie à long terme ». Ce texte est sincère il dit la vérité aux Français sur la trajectoire que nous adopterons, après une consultation qui a duré plus d'un an, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il marque, pour moi, une étape clé dans la mise en oeuvre de l'ambition du Gouvernement en matière de politique environnementale. Il poursuit un double objectif : diversification du mix énergétique, d'une part, et réaffirmation de la priorité à la lutte contre le changement climatique et à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, d'autre part.

Mes chers collègues, l'urgence climatique n'est plus à démontrer. La canicule que nous venons de traverser en a encore été la preuve. Nous devons malheureusement craindre et anticiper d'autres épisodes liés au dérèglement climatique. En octobre 2018, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié un rapport qui alerte sur les conséquences du réchauffement : montée des océans, impact important sur la biodiversité et les écosystèmes, acidification des océans ou encore risques socio-économiques majeurs, notamment pour les populations d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique centrale et du Sud. Ces témoignages, désormais quotidiens, sont le reflet d'une urgence que nous devons considérer. Le rapport est clair : nous ne pouvons contenir ce réchauffement à 1,5 degré que par des transformations radicales, en diminuant urgemment les émissions. Les catastrophes et les désastres climatiques se multiplient. À titre d'exemple, le 5 février dernier, mon collègue, Dominique Théophile, sénateur de Guadeloupe, remettait au Premier ministre un rapport sur les sargasses dans la Caraïbe. Nous le savons, la prolifération de ces algues est liée à la fois à l'élévation des températures, à l'augmentation des taux de CO2 et aux résultats des activités anthropiques. Leurs vagues successives d'arrivées, de plus en plus massives depuis 2011, représentent un véritable désastre écologique, sanitaire et économique pour les pays de la Grande Caraïbe.

Comme parlementaires, nous devons prendre notre part de l'effort : dorénavant, les futures lois de finances devront obligatoirement prendre en compte leur impact carbone et les parlementaires fixeront tous les cinq ans nos objectifs et la marche à suivre pour répondre à l'urgence.

ce texte ne renvoie donc pas uniquement à des décisions qui seront prises ultérieurement par décret. Les discussions ont été et seront encore nombreuses, et j'espère que le Sénat saura y apposer sa patte. Je vous fais confiance, mes chers collègues.

mais que, comme souvent avec le gouvernement auquel vous appartenez, nous cherchons les moyens mis sur la table pour atteindre l'objectif. La Cour des comptes européenne estime que, pour amorcer la transition écologique en France, il faudrait investir 145 milliards d'euros par an

et développer les énergies renouvelables, notamment l'éolien en mer, la méthanisation ou encore l'hydrogène décarboné ? L'urgence climatique est La COP21 de Paris s'était fixé pour objectif, en 2015, de maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Si nous ne changeons pas radicalement nos manières de consommer, de produire, de nous déplacer, notre politique énergétique et industrielle, en clair notre mode de développement, alors nous allons droit dans le mur. À cette allure, voici ce que nous allons laisser comme Terre en 2050 à nos enfants, et personne ne pourra dire que nous ne savions pas des îles englouties par la montée des eaux, des ouragans et des cyclones plus intenses, de plus en plus d'épisodes de chaleur, comme celui que nous avons connu à la fin du mois de juin, des hivers de plus en plus rudes, un million d'espèces disparues, des feux de forêt qui se multiplieront. Ce scénario n'est pas le prochain film catastrophe hollywoodien, mais la réalité en train de se préparer sous nos yeux, avec pour conséquences l'explosion de la pauvreté, avec 100 millions de pauvres en plus à l'horizon de 2030, et le déplacement de 250 millions de réfugiés climatiques à l'horizon de 2050. Bref, nous sommes en train de tuer notre planète et les espèces qu'elle porte, la nôtre incluse. Si nous ne prenons pas des décisions radicales aujourd'hui, le pouvoir politique sera devant un défi insurmontable dans dix ans comment survivre sur une planète qui a subi des dommages irréversibles, avec près de 10 milliards d'habitants ? C'est donc une politique globale et radicale qu'il nous faut mener. Ni les slogans, ni les effets d'annonce, ni la politique des petits pas ne peuvent nous sauver ! Par ailleurs, la présentation de votre projet de loi est rattrapée cruellement par l'actualité il est facile d'afficher l'objectif de la neutralité carbone en 2050 à l'article 1, mais, pendant ce temps, l'Assemblée nationale est en train de le ratifier le CETA, et l'Union européenne a signé un accord de libre-échange avec le Mercosur. Les risques sanitaires, sociaux et environnementaux sont immenses ces accords de libre-échange vont à contre-courant de l'histoire ! Alors qu'il faudrait imposer le principe de coopération entre les peuples, vous érigez le principe de compétition en dogme. Alors qu'il est urgent et vital de relocaliser notre agriculture et notre production industrielle, vous préparez treize nouveaux traités de libre-échange, qui multiplieront le transport de marchandises au-dessus de nos océans. Un jour, ces traités deviendront caducs, car ils seront reconnus comme crimes d'écocide, au même titre que les pollutions au plastique, au fioul et la déforestation à outrance pour le seul profit.

... Vous faites le pari que oui, car le capitalisme peut trouver une niche dans le développement des énergies renouvelables et réaliser des profits sur la transition verte. Cela coïncidant avec la prise de conscience de plus en plus prégnante des urgences climatiques dans l'opinion populaire, c'est tout tout un modèle de « croissance verte » qui est colporté par le Gouvernement et sa fidèle majorité. Mais, pour cela, il vous faut casser toutes les barrières, en commençant par mettre fin aux tarifs réglementés du gaz, puis en abattant progressivement les tarifs réglementés de l'électricité. Car, pour vous, une seule règle compte : la main invisible du marché ; et tant pis si cette main droite plonge des centaines de milliers de foyers supplémentaires dans la précarité énergétique ! Eh oui ! C'est ce même dogme qui vous pousse à poursuivre la vente de l'énergie nucléaire au concurrent privé d'EDF, avec le déplafonnement de l'Arenh. Là encore, alors que, contrairement à ce que vous avez affirmé, ce dispositif est, par ricochet, à l'origine de l'augmentation des tarifs réglementés de 5,9 % pour les foyers, soit près de 100 euros en moyenne, vous répondez aux injonctions des opérateurs privés et de leurs juteux profits. Pas un mot non plus sur la future concession de près de 150 barrages hydroélectriques au privé, alors qu'ils sont un élément essentiel pour stocker nos énergies renouvelables. Votre but ultime n'est pas dans la loi, mais votre plan est maintenant connu après avoir vendu Engie aux appétits financiers, vous préparez le démantèlement d'EDF. Le mécanisme est simple et connu : nationaliser les pertes, c'est-à-dire un nucléaire aujourd'hui déficitaire, et privatiser la distribution et les énergies renouvelables. Exact ! Vous voulez casser une entreprise publique intégrée pour livrer toute la filière au privé ! Mais, vous le savez, il faudra en passer par une loi pour finir de déréglementer tout le marché de l'énergie. Or, là encore, l'actualité vous rattrape, car les Françaises et les Français en ont marre de voir leur patrimoine bradé au privé, comme en témoignent les plus de 500 000 soutiens déjà exprimés au projet de loi référendaire pour Aéroports de Paris. Nous mènerons donc une bataille acharnée pour éviter le démantèlement et la privatisation d'EDF. Car,

? Répond-il à la situation d'urgence ? Même s'il est vrai qu'il comprend un certain nombre de mesures intéressantes, compte tenu des enjeux et de l'urgence, ne manquerait-il pas d'envergure ?

Mais, compte tenu du rapport du GIEC et du cri d'alarme de celui-ci, serons-nous, avec ces objectifs, sur la bonne trajectoire ? Ce texte sera-t-il compatible avec les scénarios d'un réchauffement de 1,5 degré ou avec ceux d'un réchauffement de 2 degrés, voire plus ? Étant entendu que chaque demi-degré compte.

Je ne dis pas qu'il ne comporte aucune mesure- ce ne serait ni objectif ni juste. Des dispositions sont prévues, mais qui ne répondent pas forcément aux enjeux immédiats et à l'urgence. Elles vont toutes dans le bon sens, mais le problème de ce texte que l'obligation des travaux de rénovation est repoussée en 2028, voire, pour certains immeubles, en 2033- échéances trop lointaines, assorties de trop nombreuses exceptions. Bref, l'urgence climatique est remise à plus tard, donc à très tard, peut-être même à trop tard. C'est pourquoi le groupe socialiste socialiste a présenté un amendement visant à autoriser le Gouvernement à lever un emprunt à moyen et long terme pour assurer, sans attendre, le financement des investissements dans la rénovation thermique, en aidant

je rappelle volontiers les engagements du candidat Macron pour la création d'un fonds public pour la rénovation et pour la rénovation thermique de la moitié des logements passoires en 2022.

J'y insiste, il faut une vraie politique, volontariste, dans le domaine de la rénovation, faute de quoi la France se verra accusée, comme ce fut le cas récemment, de donner volontiers des leçons, mais pas assez d'exemples. Face à des

Dans la discussion des articles, nous reviendrons sur la fermeture des centrales à charbon, sujet environnemental autant que social, et donc sur Cordemais, dont le sort était lié, selon le ministre de Rugy, au démarrage de l'EPR de Flamanville-

l'élévation de la température sous les 2 degrés, au plus près de 1,5 degré, ne relève pas de la pure convenance, sachons-le : au-delà, nous entrerions dans l'irréversible, comme le disait un ancien ministre. Je ne saurais mieux dire. Il ne s'agit pas d'en rajouter dans le registre anxiogène, mais de nous mobiliser tous et de parler vrai, sans laisser les problèmes sous le tapis.

C'est peu dire que le Parlement aura été négligé sur les sujets environnementaux depuis la récente conversion écologique du Gouvernement. Comment en effet peut-on croire un instant au respect du débat parlementaire, quand on voit le temps qui nous est laissé pour traiter de sujets aussi importants que ceux dont nous sommes Comment peut-on imaginer que le Gouvernement respecte le travail des assemblées, quand on nous propose, avec ce texte, d'avaliser une programmation pluriannuelle de l'énergie déjà rédigée depuis longtemps ? Sur ce sujet comme sur celui du Haut Conseil pour le climat, institué par décret voilà deux mois, il faudra nous expliquer, madame la secrétaire d'État, votre conception de la hiérarchie des normes

La révision des objectifs énergétiques devenait certes nécessaire, mais nous aurions pu gagner un peu de temps si les gouvernements successifs avaient davantage écouté le Sénat, qui, dès 2015, a souligné l'impossibilité objective d'une réduction de la part du nucléaire à 50 % dans notre mix en 2025.

de s'appuyer sur des points d'étape pragmatiques. Tout cela, néanmoins, ne fait pas une grande loi sur l'énergie, répondant aux défis climatiques qui sont devant nous. Où est, en effet, la « vision grand-angle » du Gouvernement sur le sujet ? Où est le dispositif courageux qui permettra de dépasser la vision punitive de l'écologie pour concilier intelligemment croissance économique, attractivité des territoires et respect de l'environnement ? Madame la secrétaire d'État, nos territoires, nos chefs d'entreprise, nos concitoyens et les élus ont besoin d'un cap clair et stable à moyen et long terme.

Le grand projet de loi Énergie-climat que nous aurions aimé voter, c'est celui qui aurait proposé une fiscalité verte positive et concilié accompagnement des ménages, progressivité de la charge et transparence dans l'utilisation des recettes. Vous choisissez de réduire la part de l'énergie nucléaire, alors que celle-ci participe aujourd'hui au bon classement de la France parmi les pays émetteurs de gaz carbonique. Et, paradoxe préoccupant, vous n'investissez que très peu dans les énergies propres ou renouvelables, en oubliant que, sans cet effort de diversification de notre mix, nous continuerons de traîner comme un boulet le solde négatif de notre facture énergétique-

collègues, ce projet de loi est décevant au regard des enjeux et des ambitions proclamées par la communication gouvernementale. Décevant par les mesures proposées, qui manquent significativement de cohérence d'ensemble,

plutôt que taxés ou montrés du doigt. Madame la secrétaire d'État, votre prédécesseur lors de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris déclarait : « L'essentiel n'est pas ce qui brille, mais ce qui dure. » Tout est dit, et chacun en mesure aujourd'hui la portée ! La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, Ronan Dantec ayant déjà pris la parole au nom du groupe du RDSE, je m'attarderai sur les mesures relatives aux passoires thermiques, qui ont fait l'objet de vifs débats aussi bien à l'Assemblée nationale qu'en commission du Sénat, la semaine dernière. Et pour cause : loin d'être anodin, le secteur du bâtiment représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre en France et dépasse largement les seuils fixés par la stratégie nationale bas-carbone, qui appelle à une rénovation thermique radicale du parc existant. Aussi, sans faire de mauvais jeu de mots, considérer qu'on peut atteindre la neutralité carbone en 2050 sans agir sur le logement, c'est aller droit dans le mur. Alors qu'un huitième des logements vendus chaque année seraient des passoires énergétiques, il y a urgence : urgence climatique, mais aussi urgence sociale. La précarité énergétique coûte cher à notre pays, et nous devons faire baisser la facture. Cet habitat énergivore recouvre plusieurs réalités réalités : des propriétaires, occupants ou bailleurs, qui ne peuvent pas se permettre de rénover leur bien ou méconnaissent les aides auxquelles ils ont droit ; parfois aussi, des marchands de sommeil qui font fortune sur l'exploitation de la vulnérabilité des occupants. La problématique n'est pas simplement urbaine elle existe tout aussi bien dans nos territoires ruraux. Il ne s'agit pas de stigmatiser ou de montrer du doigt, mais de proposer un panel de solutions adaptées à chaque situation. S'agissant des propriétaires modestes, le Gouvernement souhaite la transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en une prime unique, versée au commencement des travaux dès 2020. De notre point de vue, un meilleur accompagnement est également indispensable, car le manque d'informations lisibles sur les aides est source de nombreux renoncements. Nous proposerons donc l'ajout dans l'audit énergétique des conditions d'attribution des aides publiques et des conséquences des travaux sur la facture, la mise en place d'un parcours de rénovation énergétique parmi les missions de l'ANAH et la création dans les EPCI d'un référent chargé d'accompagner les propriétaires dans la rénovation énergétique de leur logement. En travaillant sur ce projet de loi, nous avons retrouvé deux engagements forts dans le programme du candidat Macron : l'interdiction de la location des passoires énergétiques en 2025 et la rénovation de 1 million d'entre elles d'ici à 2022. Afin d'inciter plus fermement les propriétaires qui en ont les moyens à engager des travaux, nous proposerons de définir dans la loi un seuil maximal de consommation énergétique finale des logements pouvant être considérés comme décents et de fixer un palier intermédiaire de rénovation de 1 million de logements mal isolés d'ici à 2022, conformément à l'engagement du Président de la République. Nous proposerons aussi d'instaurer sans attendre une sanction, avec l'interdiction de la location des logements classés G dès 2022 et des logements classés F dès 2028, toujours en nous inspirant des engagements du candidat Macron.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail remarquable de nos rapporteurs et de nos administrateurs, dans le contexte particulier que la présidente de notre commission a souligné. à notre examen, censé faciliter l'accès à une énergie décarbonée et abordable pour tous, se concentre sur l'offre énergétique, les tarifs et la lutte contre la fraude. Il ne s'attache pas aux sujets majeurs, tels que la maîtrise de la demande dans les secteurs les plus émetteurs et fait peu de place à l'évaluation et à l'exemplarité de l'État. En complément des observations présentées par mon collègue Jean-Pierre Moga, j'insisterai sur trois points. points. D'abord, la lutte contre le changement climatique et l'objectif de neutralité carbone. Comment atteindre zéro émission nette de carbone d'ici à 2050 en nous privant du levier des puits de carbone ? Selon des chercheurs suisses, 900 millions d'hectares de canopée en plus des 2,8 milliards d'hectares actuels pourraient absorber 205 des 300 gigatonnes de carbone rejetées dans l'atmosphère depuis la fin du XIX siècle. En ce sens, je proposerai un amendement visant à étendre le champ obligation des certificats d'économies d'énergie à la captation de carbone. En créant un volet spécifique au sein du dispositif des CEE, nous soutiendrions les investissements dans les pratiques vertueuses et les services environnementaux devenus essentiels. Je pense à tout ce qui valorise les espaces naturels et les matériaux biosourcés, préservant et développant ainsi des capacités de stockage du CO2 dans le sol et les végétaux, ainsi que des capacités de substitution par l'usage de matériaux biosourcés. autre levier : la petite hydroélectricité. Pouvons-nous véritablement nous permettre de nous priver de ce potentiel, même de petite taille ? Comment expliquerons-nous aux générations futures que, alors que notre planète étouffait, nous n'avons pas jugé nécessaire d'optimiser le potentiel d'énergies renouvelables décarbonées des petites unités Sortons du dogmatisme : les expériences des dernières années démontrent que, en matière d'énergie et de stratégie bas-carbone, il n'y a pas une solution miracle, venue des ENR électriques, mais plutôt un mix de technologies qui se complètent. sur ce sujet de l'offre énergétique, je souhaite réaffirmer la spécificité de notre pays, qui, du fait de son mix électrique essentiellement nucléaire, donc décarboné, doit rechercher d'abord une meilleure efficacité énergétique et des changements dans les usages, plutôt qu'une coûteuse conversion des moyens de production existants. Il serait opportun, madame la secrétaire d'État, de contrôler et d'évaluer la rentabilité des projets ENR, auxquels les soutiens publics devraient avoisiner 200 milliards d'euros à l'horizon de 2045. Ces soutiens massifs pèsent de plus en plus sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens et ne sont pas tenables à long terme. La CSPE explose, et 70 % de ses recettes vont désormais au soutien aux ENR plutôt qu'à la mobilité propre et à la rénovation thermique. La Cour des comptes comme la CRE appellent à un renforcement du pilotage budgétaire de ces charges et à un meilleur contrôle des appels d'offres, avec une possibilité de révision des mécanismes, notamment du fait des progrès technologiques. Le coût de la maintenance des ENR a diminué de plus 35 ces dernières années, sans que les engagements relatifs aux prix d'achat puissent être ajustés. Madame la secrétaire d'État, envisagez-vous une réflexion sur l'ensemble de la chaîne de valeur des industries ENR, au travers d'un bilan environnemental complet intégrant le transport et les matériaux, mais aussi les emplois créés ? De fait, il faut bien constater qu'il n'y a pas de développement industriel autour des ENR en France. Dans le contexte actuel d'urgence climatique, peut-on se satisfaire de stratégies qui ne permettent aucune réduction des émissions de gaz à effet de serre avant 2028 et ne mobilisent les financements que pour le remplacement des capacités de production actuelles, pourtant largement décarbonées, par de coûteuses ENR bas-carbone ?

c'est parce que l'énergie fossile a été utilisée massivement jusqu'à présent que nous faisons aujourd'hui face au péril écologique que nous connaissons sur la planète. Il appartient au Parlement de fixer les objectifs. Nous souhaitons une politique française ambitieuse en matière de réduction des gaz à effet de serre. Elle nécessitera d'accentuer le développement des énergies renouvelables et décarbonées. Cela ne doit pas nous faire oublier que la France bénéficie d'un atout considérable dans la production d'électricité décarbonée : le nucléaire,

La France doit rester en pointe sur cette technologie, en attendant que ces alternatives crédibles existent véritablement. Les énergies renouvelables doivent être encouragées des synergies doivent naître entre la production d'énergie et l'agriculture. Il est nécessaire de consolider un cadre stable et pérenne pour la filière biogaz afin de sécuriser les porteurs de projet. La production locale de méthane dispose de plusieurs avantages : elle permet une gestion des effluents agricoles, et le biogaz assure un complément de revenus aux agriculteurs et consolide la résilience de notre agriculture. L'agriculture fait déjà beaucoup pour l'environnement. Elle peut faire beaucoup aussi en matière d'énergie. Plus généralement, le couple biocarburants et agriculture est porteur de nombreuses promesses, notamment en matière de biokérosène- songeons à l'importance du transport aérien La lutte contre le changement climatique passera par nos territoires, mais aussi par le monde de l'entreprise. C'est notamment le cas pour les dispositions de lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie. Elles réaffirment notre engagement

En présentant son rapport en commission des affaires économiques, Daniel Gremillet a évoqué la pauvreté de ce projet de loi. Je partage ce constat, l'intention du texte étant essentiellement de faire entériner par le législateur les choix de la PPE. C'est donner bien peu d'importance au Parlement sur un sujet qui suscite une si grande préoccupation. Je note pour ma part deux grands absents dans les sujets qu'un texte portant sur l'énergie et le climat aurait dû aborder : l'industrie et le transport.

malgré sa qualité première en lien direct avec les objectifs du projet de loi : réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique.

sans avoir été entendus, que l'objectif de 2025 était inatteignable. La preuve en est aujourd'hui ! À quoi cela sert-il de fixer des objectifs dont on sait pertinemment qu'ils sont irréalistes ? Pour ma part, je ne suis ni pro ni anti-nucléaire, mais je salue l'excellence de la filière française, dont nous aurons forcément besoin pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Hormis le nucléaire, il y a l'industrie que l'on qualifie de lourde, celle que l'on peine à garder en France et qui a des besoins énergétiques importants. Le rapport de notre collègue Valérie Létard, présenté au nom de la mission d'information sur les enjeux de la filière sidérurgique dans la France du XXI siècle, a bien montré l'importance du coût de l'énergie pour l'industrie, notamment pour les entreprises électro-intensives. Or certaines d'entre elles verront leur contrat de fourniture historique arriver à terme en 2020, ce qui rend urgente la négociation d'un nouveau tarif, car, pour le maintien et la compétitivité de ces entreprises, des contrats de longue durée sont nécessaires. Notre collègue Jean-Pierre Vial, très investi sur ce sujet qu'il connaît bien en Savoie, a déposé un amendement en ce sens, mais il ne pourra faire l'objet d'une discussion ayant été déclaré irrecevable, bien qu'il s'agisse uniquement d'énergie Quelle est donc la réponse du Gouvernement sur ce point très important pour les entreprises industrielles fortes consommatrices d'énergie ? Le deuxième sujet que je souhaite évoquer est celui des transports, essentiellement le transport des marchandises, qui a une importance majeure pour notre économie. Ce sujet est absent du projet de loi, sous prétexte, je crois, d'en appeler à la LOM, sauf que la LOM ne l'aborde pas ! Le constat est connu depuis longtemps : 80 % des marchandises transportées le sont par la route, d'où l'engorgement des grands axes et les émissions de CO2

de l'axe Marseille-Lyon. Sur le Rhône, où la navigation est gérée par la CNR, qui par ailleurs assure la production d'hydroélectricité, le transport fluvial n'utilise qu'un tiers des capacités, alors qu'une barge poussée peut transporter en conteneurs l'équivalent de 200 à 300 camions, avec d'ailleurs un coût de transport trois fois moins important que par la route. À

Le précédent ministre de la transition écologique- je veux parler de M. Hulot-s'en était ému dans cette enceinte. L'actuelle ministre des transports s'en est elle aussi émue. Pour autant, force est de constater que rien ne bouge.

n'est ni à la hauteur des enjeux ni pourvu d'une vision globale à long terme. Nous n'y percevons pas les actions concrètes à mener face à l'urgence climatique qui s'impose à nous ni les moyens

Or de grands enjeux semblent avoir été balayés à la même vitesse que celle à laquelle nous avons dû examiner le texte, ce que je déplore à mon tour. Je pense notamment à l'absence totale des transports dans ce texte,

me conduit à une première réflexion. La diminution de la part du nucléaire introduit deux nouveautés majeures. La première est le passage d'une production d'électricité en masse, concentrée, à une production plus diffuse, répartie sur le territoire et accompagnée de la montée des énergies renouvelables, qui sont bien moins puissantes, ce qui entraîne des problèmes d'acceptabilité par nos concitoyens.

qu'il s'agisse du nucléaire ou des centrales à charbon, les plans de réemploi doivent être au coeur de ses préoccupations. Le volet social doit être pleinement inclus dans l'urgence climatique. Sur la question de la fermeture des centrales à charbon, permettez-moi de vous interroger de nouveau sur l'avenir comment maintenir le réseau dans l'ouest du pays, alors que l'EPR de Flamanville est retardé ? S'agissant de notre entreprise historique EDF, nous avons des interrogations. Sa situation est durablement fragilisée. En effet, l'essor des énergies renouvelables et les progrès en matière d'économies d'énergie peuvent entraîner à terme une chute des prix sur le marché européen, car, vous le savez, nous sommes dans le foisonnement, avec des échanges perpétuels avec nos pays voisins. Par ailleurs, le coût de production des réacteurs nucléaires d'un parc vieillissant augmente du fait d'un taux d'utilisation en baisse, de la multiplication des arrêts, du grand carénage qui se met en place et des problèmes de sécheresse dus au réchauffement climatique. À cela s'ajoutent les obligations de l'Arenh. L'intérêt stratégique doit être au centre de la résolution de cette équation. Le groupe socialiste et républicain attend de ces débats des avancées sur les dispositions que nous jugeons insuffisantes : la rénovation thermique et l'incitation à la mobilité verte, afin de diminuer drastiquement notre empreinte carbone. Nous devons opter pour des comportements plus sobres et plus vertueux. Afin d'assurer une continuité du service public et des politiques en faveur de l'intérêt général qui lient urgence écologique et responsabilité sociale, nous défendrons des propositions très concrètes pour lutter contre la précarité énergétique qui touche un trop grand nombre de nos concitoyens. Enfin, la lutte contre le réchauffement climatique est liée aux écosystèmes. Nous nous étonnons que nos amendements sur la préservation de la biodiversité aient été déclarés irrecevables.

tous plus ambitieux les uns que les autres sans les assortir des moyens nécessaires à leur réalisation. Pis, il se contente de ces objectifs à long terme, sans dire concrètement comment mettre en oeuvre, demain matin, des dispositifs pour une véritable transition énergétique dans les territoires. À ce titre, le projet de loi est décevant. Il manque singulièrement d'envergure et, surtout, de traduction effective de proclamations politiques pourtant largement déployées à l'article 1 à grand renfort de dates, d'estimations diverses et de calculs qui m'impressionnent neutralité carbone pour 2050, facteur 6 pour les émissions de gaz à effets de serre, réduction de la consommation des énergies fossiles à 40 %, production d'énergie hydraulique à 27 gigawatts en 2028 ou encore 40 % d'hydrogène bas-carbone dans la consommation industrielle En vérité, je me demande sincèrement si tout cela est bien sérieux ... C'est vrai ! ... et s'il ne s'agit pas simplement de servir la cause d'une diminution significative de la production nucléaire dans notre pays, mesure idéologique prise durant le précédent quinquennat

En inscrivant l'urgence écologique et climatique dans ce texte, chacun comprend qu'il faut aller vite pour réduire nos émissions de CO2. Alors pourquoi renoncer à la production nucléaire, la plus vertueuse dans ce domaine ? Réduire à 50 % la part de notre production d'électricité d'origine nucléaire ne restera qu'une annonce idéologique sans un plan d'action concret de diversification de notre mix énergétique. Bravo ! Dans ce contexte, pourquoi ne pas privilégier davantage l'hydrogène, Chacun sait qu'on ne progresse pas parce qu'on a peur mais parce qu'on croit au progrès. Pour paraphraser le cheikh Yamani, « l'âge de pierre ne s'est pas arrêté faute de pierres Je veux poursuivre mon propos en évoquant la rénovation énergétique des logements, sujet ô combien important, puisque le bâtiment représente environ 45 % de la consommation d'énergie dans notre pays. pays. Si les objectifs affichés depuis plusieurs années semblent volontaristes, autour de 500 000 logements rénovés par an, on est loin d'une mise en oeuvre effective et unifiée sur le terrain. J'en veux pour preuve le caractère très flou des missions du service public de la performance énergétique de l'habitat. Pourtant, tous ceux qui ont une expérience dans ce domaine peuvent témoigner de la nécessité de clarifier le jeu des nombreux acteurs, de faciliter l'accès à un conseil neutre, indépendant et efficace pour les particuliers, déboussolés par la multitude des messages auxquels ils sont régulièrement confrontés. Une stratégie globale est à arrêter, avec sans doute les régions comme chefs d'orchestre et- pourquoi pas ?-les intercommunalités comme relais dans les territoires. Vous le savez, madame la secrétaire d'État, la rénovation thermique d'un logement peut être onéreuse- elle coûte 30 000 euros en moyenne, et parfois bien plus. Cela mérite de concentrer nos efforts sur cet axe. Sur le sujet de ce qu'on appelle les passoires énergétiques- on en dénombre environ 7 millions dans notre pays -, nous devons faire preuve d'imagination, non pas pour sanctionner et taxer toujours plus, mais au contraire pour encourager et valoriser les propriétaires bailleurs qui effectuent les travaux. Je proposerai un amendement en ce sens.

qui conçoit que des changements de comportement et des efforts de rénovation vont être nécessaires, mais qui aspire à une déclinaison pragmatique expurgée de toute empreinte idéologique. La parole

De plus, tout ne se décide pas au niveau national, tout ne dépend pas de l'État. Il peut tout de même ! Les collectivités territoriales sont aussi des acteurs importants. Vous l'avez dit, la mobilisation territoriale est absolument essentielle. Je travaille avec les collectivités territoriales depuis que j'ai reçu le portefeuille de secrétaire d'État au ministère de la transition écologique et solidaire. Nous travaillons pour le déploiement de la transition écologique et solidaire au quotidien au plus près des territoires. Les collectivités territoriales auront à apporter une partie de la réponse aux questions qui nous sont posées : la rénovation des bâtiments, les transports, le développement des énergies renouvelables. Vous avez parlé de l'industrie.

Nous devons porter attention aux plus modestes, à ceux qui sont touchés de plein fouet par le changement climatique, aux ménages dont le budget ne permet pas de faire face à l'augmentation des factures. C'est important, car notre modèle social est en cause.

c'est un maillon d'un système qui va nous permettre d'aller plus vite, plus fort et d'atteindre les objectifs que nous nous fixons en matière de transition écologique. Ces objectifs sont-ils compatibles avec l'accord de Paris ? La réponse est oui ! Ils sont compatibles

l'accompagnement est en place. Nous avons pris l'engagement de fermer ces centrales d'ici à 2022. Cet engagement sera tenu en respectant la sécurité d'approvisionnement. Les scenarii réalisés par RTE

revenir au système qui existait avant 2017 et trouver la base juridique permettant de définir le rôle du préfet de manière équilibrée, de sorte que l'autorité environnementale puisse rendre des avis et que les projets puissent être mis en oeuvre. Nous ne démantelons donc pas du tout l'autorité environnementale.

mais aussi pour le Parlement, qui disposent tous deux du pouvoir de ratifier les traités dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution. En second lieu, l'étude préalable à la ratification d'un accord, quand bien même elle présenterait des gages d'indépendance, sera toujours sujette à caution. Pour s'en convaincre, il suffit de se souvenir de l'étude élaborée à la demande du Gouvernement sur l'accord de libre-échange avec le Dans ce contexte, le dispositif proposé pourrait ne pas suffire à introduire davantage de rationalité dans les choix de politique internationale. Enfin et surtout, il n'est pas besoin d'empêcher la ratification d'un accord contraire aux engagements internationaux et européens de la France en matière d'énergie et de climat. En effet, ces engagements sont pleinement applicables, et la France ne saurait les dénoncer pour leur préférer des engagements de sens contraire. La commission a donc émis un avis défavorable

Nous nous attacherons aussi à évaluer pleinement les effets de l'accord avec le Mercosur, qui, lui, n'est pas encore entré en vigueur et n'entrera en vigueur qu'après une décision à l'unanimité du Conseil européen. Ce n'est pas la peine d'inscrire le principe de cette expertise indépendante dans la loi, puisqu'elle est déjà mise en oeuvre. De plus, la formulation retenue dans le dispositif de l'amendement est très générale et a relativement peu de portée pratique, car il est quasiment impossible de déterminer si un accord en particulier

ni les textes finaux, ni les études d'impact que vous évoquez. Si vous les avez, rendez les publics ! Organisez de grands débats sur les chaînes audiovisuelles publiques, afin de mettre

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Merci